Madame la présidente,

pourtant nécessaire pour aborder des questions aussi épineuses. C'est pourquoi la commission des lois s'est montrée ouverte aux seuls amendements qui ne concernaient pas des questions dont la complexité appelait des débats approfondis. Sous réserve de précisions rédactionnelles et d'un report à 2018 de l'application de ces modifications, la commission des lois a suivi mes propositions et adopté le texte tel qu'il vous est présenté,

La réelle innovation de cette proposition de loi est d'obliger les partis politiques à faire figurer en annexe de leurs comptes les informations relatives aux emprunts souscrits et consentis. Alain Anziani a ainsi fait référence à l'emprunt russe souscrit par un parti d'extrême droite. Ces informations seraient soumises à la certification des commissaires aux comptes chargés d'examiner actuellement les comptes déposés auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Cette dernière disposerait ainsi d'informations vérifiées sur ce point. Je rappelle que ce type d'informations est déjà transmis à la Commission nationale des comptes de campagne par les candidats, au travers de l'annexe n° 3 au compte de campagne.

Il s'agit en réalité de la généralisation d'une publicité qui est déjà possible sur demande d'un tiers, dès lors que les documents reçus par la Commission nationale des comptes de campagne sont considérés comme des documents administratifs, communicables à toute personne.

un doute, que j'avais exprimé en commission la semaine dernière, sur l'étendue des informations à transmettre et publier en matière de flux financiers entre partis politiques : un amendement : un amendement de François Pillet nous permettra de revenir précisément sur cette question. Ce texte accompagne un effort de transparence financière, qui recueille un large assentiment. Qui pourrait s'y opposer

et républicain, vise à modifier le code électoral et la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique pour renforcer la transparence des relations financières existant entre les candidats aux élections politiques, les partis et les acteurs économiques et financiers.

pour donner automatiquement les moyens à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de vérifier la légalité de ces financements. Ce texte poursuit également l'objectif d'informer les citoyens pour leur permettre d'apprécier par eux-mêmes l'influence que ces relations pourraient avoir sur l'indépendance des formations et des candidats. La proposition de loi vise, enfin, à étendre l'obligation de la communication et de la publication aux flux financiers entre les partis, et entre les partis et les candidats, puisqu'un parti peut lui-même souscrire un emprunt et en transférer le bénéfice du capital à son candidat. En outre, ce texte répond à l'enjeu global de transparence financière de la vie politique sur lequel le Gouvernement s'est engagé, depuis 2012, à travers la mise en place de nouveaux mécanismes de publicité et de contrôle. Il s'inscrit d'abord dans le prolongement des lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique, qui ont marqué une avancée significative- chacun le reconnaît -en termes de respect de règles éthiques par les responsables publics, avec notamment l'obligation faite aux parlementaires et aux membres du Gouvernement de publier leurs déclarations d'intérêts et de patrimoine. Il reprend ensuite les termes de l'article 30 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, que le Conseil constitutionnel avait censuré pour des raisons de procédure législative. Enfin, la proposition de loi contribue, de manière équilibrée, au respect de principes et d'objectifs de valeur constitutionnelle indispensables à la vie démocratique de notre nation. Elle conforte le droit des acteurs politiques à recourir à l'emprunt. De surcroît, en ne s'imposant qu'aux partis politiques bénéficiaires de l'aide publique et qui choisissent donc librement de se soumettre aux dispositions de la loi de 1988, elle s'inscrit dans le respect du principe de liberté de formation et d'activité des partis politiques consacré par l'article 4 de notre loi fondamentale. De plus, en fixant des critères clairs, objectifs et identiques pour l'ensemble des partis politiques, la proposition de loi assure le respect des principes d'égalité et de pluralisme des opinions, qui constituent le fondement de la démocratie. Concernant son application, la commission des lois a opportunément adopté un amendement du rapporteur prévoyant une entrée en vigueur différée de ces dispositions, qui seront donc applicables aux élections se déroulant après le 1 janvier 2018 et aux comptes arrêtés au titre de l'exercice 2018.

qui devront déposer leurs comptes au titre de l'exercice 2016 ne seront pas modifiées. Quant à l'application de cette proposition de loi aux élections présidentielles ultérieures, elle ne sera envisageable qu'à la condition de modifier l'article 4 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, modification qui n'est possible que par une loi organique. Partant de ce constat, le Gouvernement est favorable au renforcement des obligations comptables des partis politiques. Il contribuera à réaliser le double impératif démocratique d'exemplarité des acteurs politiques et d'information des citoyens,

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, cette proposition de loi d'Alain Anziani est particulièrement opportune.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, cette proposition de loi, feutrée, discrète, sans envergure apparente, soulève à mon avis de grandes questions qui dépassent le cadre étroit d'aujourd'hui. En premier lieu, se posent des questions de forme, d'opportunité : pourquoi ce texte vient-il en débat aujourd'hui ou, plutôt, pourquoi seulement aujourd'hui ? Pourquoi est-il porté par un parlementaire et un groupe ? Pourquoi le Gouvernement ne s'en est-il pas saisi ? Pourquoi le Conseil Constitutionnel a-t-il censuré une telle disposition qui, de toute évidence, avait sa place dans la loi Sapin II ? Quelle est la légitimité du Conseil constitutionnel à censurer à tour de bras des dispositions votées par les représentants du peuple, comme à l'occasion du dernier texte relatif à l'égalité et à la citoyenneté, dont 36 articles- pas moins ! -ont été balayés par les juges du Palais-Royal ? de loi peut-elle répondre un seul instant à la grande attente de nos concitoyennes et concitoyens en matière de refondation politique ? avez-vous conscience que nous débattons aujourd'hui au Sénat d'un texte relatif aux obligations des partis et candidats en matière de financement, alors que notre pays est, une fois de plus, une fois de trop peut-être, traversé par une polémique de grande envergure sur des malversations supposées

répond-elle un seul instant aux interrogations, à la colère du peuple ? Je le dis franchement, mes chers collègues, discuter de cette question fondamentale des rapports entre l'argent et la politique dans ces conditions, ici, au Sénat, ne relève-t-il pas pas d'une provocation ou, au minimum, d'une grande maladresse, sans doute involontaire, à l'égard du peuple ? Serions-nous, seriez-vous, à ce point coupés de la réalité pour ne pas voir cela ? Nos concitoyens veulent une transparence totale quand l'argent public est mêlé à la vie politique. Ils veulent la probité, car leur vie est dure : depuis des années, des décennies, on leur demande de se serrer la ceinture, de payer des impôts pour régler les difficultés du pays. Ils ne supportent plus de constater les détournements d'argent public ou les pratiques frauduleuses commis par ceux qu'ils ont mandatés pour gouverner, pour les représenter. Le texte qui nous est soumis concerne principalement la transparence, la publicité et l'inscription dans les comptes des emprunts contractés par des partis ou groupements politiques, ou par des candidats, même si l'intitulé du texte initial n'évoquait pas ces derniers. Selon le rapporteur lui-même, cette proposition de loi a pour origine un amendement du groupe socialiste déposé à l'Assemblée nationale à l'occasion de l'examen du texte dit Sapin II relatif à la lutte contre la corruption, qui, je l'ai dit, fut retoqué par le Conseil constitutionnel comme étant un cavalier législatif motif qui, personnellement, m'échappe quelque peu ... Cette proposition de loi vise donc, selon M. le rapporteur, les emprunts russes contractés par le Front national, dont le montant pourrait être de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il y a donc matière à à légiférer, c'est une évidence, même si l'exclusion des emprunts auprès de personnes physiques est prévue, ce qui peut paraître dommageable lorsque l'on sait que certains candidats, pour ne pas en viser un plus précisément, organisent des repas à la à plus de 7 000 euros le couvert Ne faudrait-il pas une certaine publicité des dons ou emprunts concernant des personnes physiques au-delà d'un certain seuil ? La volonté de transparence des auteurs de la proposition de loi les

à six mois la période de comptabilisation des dépenses de campagne ? Comment peut-on raisonnablement porter l'idée d'assainir les relations entre argent et politique en poussant objectivement à la hausse des dépenses de campagne, puisque le plafond de ces dernières n'a pas été réduit proportionnellement à la réduction d'un délai d'établissement des comptes de campagne ? Cet appel d'air à dépenser davantage est en contradiction avec l'esprit qui anime la présente proposition de loi. Notre groupe, quant à lui, porte l'idée d'une réduction forte du plafond de dépenses de campagne autorisé. Je l'ai donc dit d'emblée, ce texte m'interroge,

Pourquoi ne pas avoir déposé une proposition de loi organique simultanément ? La mesure adoptée en commission de reporter à 2018 l'application du texte est vraiment surprenante.

mais il ne fallait pas présenter ce texte pour renoncer à l'appliquer immédiatement. C'est notre sentiment, car l'opinion publique y verra une nouvelle fois des intentions inavouables, alors que- j'en suis persuadée -ce n'est pas le cas. Nous proposerons donc un amendement pour rétablir le texte d'origine sur la question des délais, car nous ne pouvons cautionner un coup d'épée dans l'eau. Au regard de cet affichage et de l'absence de démarche audacieuse et globale en matière de transparence, au regard de l'adoption récente de la réduction du délai pris en compte pour l'établissement des comptes de campagne, le groupe CRC ne peut voter en l'état cette proposition de loi ; il s'abstiendra. La parole

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, ces dernières années, nous avons eu de multiples occasions de débattre des moyens de restaurer la confiance de nos concitoyens dans leurs institutions et de la nécessité de « moraliser » la vie publique. Depuis 1988, la France s'est dotée d'un arsenal législatif parmi les plus rigoureux au monde au regard des critères érigés par l'OCDE. Durant ce quinquennat, une énergie considérable a été mobilisée pour ériger l'impératif de transparence à un rang quasi constitutionnel, s'imposant à la vie économique comme à la vie publique. Il faut faire attention toutefois aux effets pervers : trop de transparence ne peut-elle pas nuire à la transparence ou, du moins, à une vie démocratique sereine et apaisée ? Car on n'ira jamais assez loin dans la transparence et, dans ce cas, nous ne ferons qu'accroître la défiance envers les élus de la République ! Malgré toute l'énergie déployée ces dernières années, on constate que la construction de ces nouvelles normes n'a eu qu'un effet relatif sur la perception de la corruption par nos concitoyens. Si l'on analyse les travaux de l'organisation Transparency International, souvent présentée en référence par les défenseurs de la cause, cette perception s'est faiblement améliorée entre 2015 et 2016 et a stagné entre 2016 et 2017. Il faut donc s'interroger sur les effets réels de ces textes sur nos relations avec nos concitoyens. Jusqu'à présent, le principe de transparence joue comme une présomption d'improbité contre ceux qui y sont soumis, dont la valeur serait supérieure à celle de la présomption d'innocence. Il en va de même pour la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui : la publication de l'identité et de la nationalité des établissements bancaires consentant des prêts aux formations politiques et aux candidats sans intermédiation d'un juge apportera-t-elle une information utile à nos concitoyens ? Quelle vérité révèle-t-elle de l'intention et de la sincérité d'une formation politique ? Au contraire, cette proposition de loi méconnaît la réalité du financement de notre vie politique. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ainsi que le Conseil constitutionnel ont déjà accès à un nombre considérable de documents permettant de vérifier la provenance des financements des partis politiques et des candidats. En 1995, le Conseil constitutionnel avait par exemple requalifié un emprunt contracté par le candidat Balladur dans son compte de campagne. Ces éléments font également déjà l'objet d'une publication. En raison des différentes règles encadrant déjà les moyens de financement des partis politiques, on sait que ceux-ci sont aujourd'hui principalement financés par l'aide publique qui leur est versée, en fonction de leur poids aux élections et au Parlement. Nous le savons, ce mécanisme a pour effet de renforcer les grandes formations.

des sources de financement des candidats à l'élection présidentielle sont de 47 % pour l'apport personnel, contre 26 % pour les dons des personnes physiques et 25 % pour la contribution des partis. Il faut en déduire que le recours à l'emprunt est devenu incontournable pour financer la participation de candidats aux campagnes électorales, pour les petites formations politiques ou pour les formations nouvelles qui ne disposent pas du concours des aides publiques. En outre, comme cela a été largement médiatisé, le rejet des comptes de campagne du président sortant en 2012 a créé un précédent les banques, qui prennent désormais en compte cet aléa moral, se montrent beaucoup plus réticentes à accorder des prêts aux candidats. Les présidents de la Société Générale, de LCL, du Crédit mutuel ou encore de HSBC se sont clairement positionnés sont clairement positionnés sur le sujet. Dans ce contexte, il est à craindre que ces nouvelles exigences de transparence constituent un nouveau facteur de découragement des établissements de crédit. À terme, cette proposition de loi pourrait empêcher les petites formations politiques et les formations nouvelles de présenter des candidats aux élections, et donc s'ériger comme un obstacle à la représentativité. C'est totalement contraire à ce que nous défendons et incarnons au sein de notre groupe nous sommes pour la prise en compte de la diversité des sensibilités politiques, car elles font la richesse de notre vie démocratique ; nous sommes contre le dualisme partisan, toujours artificiel et résultant de règles institutionnelles avantageuses pour les deux grands partis. Mes chers collègues, la défiance des Français envers notre vie politique vient aussi beaucoup de là : la bipolarisation accrue et le dualisme partisan, qui verrouille le débat et empêche la construction de majorités d'idées Soyons modernes ! Dépassons le vieux clivage droite-gauche, devenu totalement inopérant ! Enfin, j'ajoute qu'au-delà de nos interrogations sur la pertinence à publier de manière indiscriminée des données à valeur informationnelle variable, dans le seul but de restaurer la confiance de nos concitoyens dans nos institutions démocratiques, cette proposition de loi pose également la question de l'équilibre à établir entre le principe de transparence et celui de représentativité. Quel intérêt y aurait-il à accroître la transparence du fonctionnement de notre démocratie représentative si le principe représentatif n'était pas matériellement garanti ? En conséquence, les membres du groupe du RDSE n'approuveront pas cette proposition de loi, qui, une nouvelle fois, sous un intitulé séduisant,

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues,

informer le plus possible sur les emprunts que les forces politiques sont amenées à contracter pour mener leur action politique ; veiller aux transferts entre

De plus, ces mesures viennent combler un vide juridique, ce qui va dans le bon sens. Il s'agit d'imposer davantage d'obligations comptables aux partis politiques et aux candidats concernant notamment leurs emprunts bancaires, mais également d'apporter à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques des données explicitant ces relations financières et de lui donner les moyens de vérifier leur légalité.

ou la cessation des fonctions du mandataire financier d'une campagne électorale sur celui applicable aux décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui est de six mois. Cela permettra notamment aux candidats de connaître le montant exact de l'éventuelle dévolution. Il s'agit là d'une recommandation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Jean-Pierre Grand. Cet amendement vise à permettre à un candidat d'effectuer une dévolution au profit d'un mandataire financier d'un parti politique, possibilité aujourd'hui uniquement réservée au profit des associations de financement des partis politiques. Il s'agit là également d'une recommandation de la Commission nationale

En effet, en perdant le bénéfice de certaines dispositions de la loi du 11 mars 1988, un parti politique redevient une personne morale de droit commun. II s'agit là de codifier une jurisprudence du Conseil d'État. Quel est l'avis de

Actuellement, parmi les personnes morales, seul un parti politique peut soutenir financièrement un candidat. Si un parti ne respecte pas ses obligations comptables, il n'est plus considéré par le juge comme un parti politique.

Le droit actuel relève d'un pur constat et ne procède pas d'une logique punitive, qui induit une procédure quasi juridictionnelle pour la prononcer, ouvrant également des recours contre cette décision.

Jean-Pierre Grand. Cet amendement vise à compléter les mentions obligatoires devant figurer sur les documents d'appel aux dons des candidats dans le cadre de leur campagne électorale, en y ajoutant le plafond maximal de 4 600 euros,

votée en 2011. En effet, en l'état actuel de nos finances publiques, les candidats doivent faire preuve de modération. Il conviendra d'adopter une loi organique pour appliquer cette baisse à l'élection présidentielle.

sous réserve de dispositions spécifiques pour les élections sénatoriales, au chapitre V du titre I du livre I du code électoral. Au sein de ce chapitre, le dernier alinéa de l'article L. 52-11 prévoit depuis 2011 un gel temporaire des plafonds des dépenses électorales. Ce gel s'applique donc aux élections sénatoriales. L'adoption de cet amendement pourrait d'ailleurs conduire à un raisonnement et à exempter ainsi nos collègues sénateurs représentant les Français établis hors de France de ce gel, car l'amendement ne vise pas à reproduire cette disposition au sein l'article 48 de la loi du 22 juillet 2013, qui s'applique à leur élection. Or je n'imagine pas un seul instant que vous ayez envisagé, mon cher collègue,

le plafond annuel maximal de 7 500 euros, l'interdiction du financement par les personnes morales et les sanctions encourues en cas de violation de ces dispositions. Il s'agit d'un droit légitime à l'information des personnes physiques cotisantes ou donatrices et permettant notamment d'éviter les dépassements accidentels de plafond. Il s'agit, là aussi, d'une recommandation de la Commission nationale Monsieur le rapporteur,

amendement vise à supprimer l'actualisation annuelle par décret de certains montants relatifs aux dons aux partis politiques. En sus du gel actuel des actualisations, cette suppression permet de rétablir une peine contraventionnelle, accidentellement abrogée en 2011, prévue en cas de violation des obligations d'information. Il s'agit, là encore, d'une recommandation de la Commission nationale des comptes de campagne.

En deçà de ce seuil, la certification par un seul commissaire aux comptes apporterait toujours des garanties suffisantes et permettrait d'alléger la charge financière pesant de fait sur ces partis de moindre envergure. Il s'agit de nouveau d'une recommandation de la Commission nationale

Grand. Le présent amendement vise à instaurer une obligation de rotation des commissaires aux comptes des partis politiques, en limitant leur mandat à six exercices consécutifs. Une telle obligation existe déjà dans le code de commerce pour les associations faisant appel public à la générosité. Là encore, il s'agit d'une recommandation de la Commission nationale

du constat et ses conséquences juridiques. Aujourd'hui, tout non-respect des obligations comptables entraîne la perte du bénéfice de certaines dispositions, les fractions des aides publiques par exemple, et de la possibilité de délivrer des reçus de dons pour déduction fiscale

? Le Gouvernement n'est pas opposé par principe à une réflexion de fond sur l'évolution des pouvoirs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, afin notamment d'adapter, comme vous l'indiquez, les

Jean-Pierre Grand. Sans remettre en cause la liberté constitutionnelle de création et d'organisation des partis politiques, je propose, au travers de cet amendement, d'interdire à un parti politique sanctionné pour non-respect de ses obligations comptables de recevoir des contributions financières d'autres partis politiques. Une formation politique défaillante peut créer un parti politique frère dans l'unique but de se substituer à elle l'année suivante pour l'encaissement des dons et cotisations. Ensuite, en toute légalité, ce nouveau parti peut lui reverser les fonds, rendant ainsi inopérante la sanction prononcée. Il s'agit d'une autre recommandation de la Commission nationale Monsieur le rapporteur,

Monsieur le rapporteur,

adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre

vous apprêtez à examiner une proposition de loi dont l'initiative revient à votre collègue député, le Lorrain Dominique Potier. Ce texte poursuit plusieurs objectifs que partage le Gouvernement il est fidèle aux valeurs humanistes qui fondent notre République ; il est le reflet de l'attention que les femmes et les hommes de progrès accordent à la protection des droits fondamentaux et de notre environnement. La mondialisation est une réalité. Il ne s'agit pas de la combattre, mais de l'encadrer, afin qu'elle ne tourne pas à l'exploitation sans retenue, hors de notre territoire, des personnes et de l'environnement. Cette proposition de loi est tout sauf un texte de circonstance, rédigé à la hâte. Le texte qui vous est présenté aujourd'hui est le fruit d'une large concertation d'échanges nourris avec la société civile, en particulier les ONG. Son ambition est de porter à un très haut niveau le devoir de vigilance des entreprises en matière de protection des personnes et de l'environnement. C'est pourquoi, depuis son examen en première lecture, le Gouvernement soutient cette proposition de loi fidèle aux valeurs qu'il a toujours défendues et cherché à promouvoir. L'idée de responsabiliser les très grandes entreprises en raison de leurs activités à l'étranger n'est pas une nouveauté. Elle traverse le débat public depuis le début des années 2000, au niveau tant national qu'européen et international. À l'échelle nationale, notre gouvernement, dans le sillage des engagements pris par le Président de la République, a oeuvré en ce sens par l'adoption des lois du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative relative à la politique de développement et de solidarité internationale et du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, plus connue sous le nom de loi Sapin II. Ce n'est qu'un début. Nous continuons de travailler en faveur de la transparence et d'une économie plus respectueuse des valeurs fondatrices de notre société dans le cadre de la transposition de la directive européenne du 22 octobre 2014 la responsabilité sociale et environnementale. Permettez-moi, à ce sujet, de rappeler que le texte qui vous est présenté aujourd'hui n'a pas vocation à transposer cette directive. C'est dommage ! Ses objectifs sont autres, bien qu'il s'inscrive dans le même mouvement de fond. L'esprit de la proposition de loi n'est pas inconnu. Il relève des mêmes principes que ceux qui ont guidé et continuent de guider notre action en matière de prévention de la corruption dans le monde économique. Pourtant, mesdames, messieurs les sénateurs, il semblerait, si je saisis bien les intentions de la majorité sénatoriale, que vous allez faire le choix de ne pas débattre de ce texte, auquel, par posture, vous aviez déjà réservé un fort mauvais accueil en première lecture. L'observateur attentif ne pourra que s'en étonner. Tout d'abord, vous avez fait vôtre la philosophie de ce texte lors de l'examen de la loi Sapin II, sans que cela heurte votre sensibilité. La proposition de loi étend cette obligation de vigilance, selon des modalités différentes, mais dans un même esprit, aux atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales dans les domaines de la santé, de la sécurité des personnes et de la protection de l'environnement. Qu'y a-t-il de condamnable dans cette entreprise ? Ensuite, le texte soumis à votre commission des lois a évolué positivement depuis le premier examen que vous en avez fait en 2015. La nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, en lien avec le Gouvernement, a permis d'en préciser la rédaction dans l'objectif d'accroître la sécurité juridique du dispositif. Ainsi, l'article 1 a été amendé pour fixer la liste des mesures de vigilance qui devront être appliquées par les entreprises. Cet ajout permet de guider ces dernières dans la mise en oeuvre des nouvelles obligations qui leur incombent. Ont également été précisées par l'Assemblée nationale les conditions dans lesquelles la responsabilité civile des entreprises pourra être engagée en cas de manquement à l'une de leurs obligations de vigilance. En outre, a été ajoutée l'obligation de mettre en demeure, préalablement à la saisine du juge, la société en cause afin qu'elle se mette en conformité avec ses devoirs de vigilance. Enfin, la proposition de loi a été complétée par un article 4, lequel, inspiré par vos travaux lors de la deuxième lecture, prévoit l'application dans le temps du dispositif pour permettre aux entreprises de remplir convenablement leurs obligations après l'entrée en vigueur de la loi. Toutes les conditions sont réunies pour poursuivre ce travail de précision rédactionnelle afin d'améliorer l'efficacité juridique du texte et de garantir sa mise en oeuvre dans les meilleures conditions. Il aurait été possible de trouver des solutions d'équilibre pour aboutir à un compromis dont chacun aurait pu être fier. Fier de soutenir une proposition de loi qui combat les dérives de la mondialisation. N'y a-t-il pas, en effet, une forme d'hypocrisie à considérer que nos entreprises n'ont à être vertueuses qu'à l'intérieur de nos frontières nationales ou européennes ? Or je crains de devoir bientôt constater le rejet de ce texte par la majorité sénatoriale. L'occasion vous était pourtant donnée, mesdames, messieurs de l'opposition, d'en parfaire la rédaction. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous nous avez accoutumés à ces barouds d'honneur. Je ne reviendrai pas ici sur les entraves que vous avez posées au débat démocratique

tout comme l'échec récent de la commission mixte paritaire, pourraient laisser penser que les drames sur les sites de production à l'étranger ou que la dégradation de notre environnement vous laissent insensibles. Ces préoccupations devraient nous rassembler. Par-delà les clivages partisans, elles visent l'intérêt général, à l'échelle tant nationale que planétaire. Vous faites le choix d'occulter la mobilisation de la société civile et le travail parlementaire considérable réalisé depuis de longs mois. Le Gouvernement, les organisations non gouvernementales, syndicales et patronales ont oeuvré de concert pour bâtir ce texte. Et vous ne trouvez rien de mieux que de lui opposer une fin de non-recevoir Vous affirmez, sans le démontrer, que ce texte portera atteinte au développement et au dynamisme de notre tissu productif. Bien sûr, il n'en est rien ! Ce gouvernement n'a pourtant cessé d'oeuvrer en faveur de la compétitivité de nos entreprises. Comment imaginer aujourd'hui qu'il veuille lui nuire ? Mais, comme il n'est pas indifférent à la régulation éthique de la sphère économique, le Gouvernement souhaite que cette proposition de loi soit adoptée par le Parlement et appliquée dans les meilleurs délais. Mesdames, messieurs les sénateurs, le travail parlementaire aurait pu, aurait dû, se poursuivre. Le Gouvernement avait exprimé, lors de l'examen à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, des réserves sur certains points du texte au regard de la Constitution. Il avait, à ce titre, titre, insisté sur la nécessité de l'ajuster, notamment en matière de proportionnalité des sanctions. Cependant, votre lecture partisane de cette proposition de loi a bloqué toute possibilité d'approfondir le travail parlementaire. Cette posture a de quoi indigner nos concitoyens, qui attachent une grande importance à la défense des droits fondamentaux et à la protection de l'environnement. Le temps est révolu où les multinationales pouvaient poursuivre leurs activités et réaliser des profits sans se soucier des conditions dans lesquelles elles travaillaient. Les scandales les plus récents l'ont montré : les entreprises coupables de mauvais comportements voient leur image ternie par de tels événements. L'entrée en vigueur de ce texte préviendra de tels comportements dans l'intérêt de tous et évitera que les grands groupes n'abîment leur image par négligence- une négligence d'une autre époque que nous devons combattre sans relâche pour continuer de bâtir un monde plus juste et plus responsable. Ce sont nos concitoyens eux-mêmes qui l'exigent ! C'est pourquoi, aux côtés de ses auteurs, nous pensons que cette proposition de loi est utile et fidèle aux engagements du Gouvernement en faveur de la responsabilité des entreprises.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous sommes saisis en nouvelle lecture du texte de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, et ce, pour la troisième fois Nous avions pourtant, en deuxième lecture, fait des pas vers nos collègues députés en proposant de transposer une partie des obligations en matière de vigilance prévues par la directive de 2014 sur la publication d'informations non financières par les grandes entreprises. Nous n'avons, hélas ! pas convaincu les députés, et la commission mixte paritaire a échoué. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a réécrit son texte, mais en conservant son approche punitive de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Ce n'est pas la nôtre. Et cette nouvelle version du texte ne répond que très partiellement aux objections du Sénat En première lecture, tout en souscrivant à l'objectif qu'elle poursuit, le Sénat avait rejeté la proposition de loi en raison des incertitudes juridiques, notamment constitutionnelles, et des risques économiques d'atteinte disproportionnée à la compétitivité des entreprises françaises et à l'attractivité de la France. Il avait considéré que le niveau pertinent pour traiter d'une telle problématique était celui de l'Union européenne. Contrairement à ce qui s'était passé en deuxième lecture, la position des députés en nouvelle lecture a évolué, mais pas suffisamment pour répondre à nos critiques économiques et juridiques. Les problèmes de nature économique et pratique soulevés par le principe même de cette proposition de loi demeurent entiers. Une des difficultés constitutionnelles exprimées en première lecture a bien été prise en compte par nos collègues députés, au regard du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. L'Assemblée nationale a ainsi précisé le contenu du plan, c'est-à-dire le contenu de l'obligation sanctionnée par une amende civile et un régime spécifique de responsabilité. Le Sénat avait relevé l'incertitude entourant les normes de référence sur la base desquelles le plan de vigilance devait être élaboré, rendant incertain le contenu même de l'obligation, alors que des sanctions seraient encourues en cas de manquement à cette même obligation. Une telle incertitude soulevait une difficulté réelle au regard du principe de légalité des délits et des peines. Outre la finalité générale du plan de vigilance, la proposition de loi précise désormais la nature de ces mesures, même si un décret en Conseil d'État peut en compléter la liste, ce qui soulève à nouveau une difficulté au regard du principe de légalité des délits et des peines. Le texte précise désormais- utilement -que les filiales et les sociétés contrôlées dépassant les seuils sont réputées remplir leur obligation de vigilance si la société mère met en place un plan de vigilance qui les englobe. Cela ne doit cependant pas conduire à une ingérence irrégulière de la société mère dans la direction et la gestion de ses filiales et sociétés contrôlées. Dans un souci de simplification qui doit être salué, la prévention de la corruption n'est plus abordée dans le cadre du plan de vigilance, par coordination avec l'obligation de mettre en place des mesures destinées à prévenir et à détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence, déjà instaurée, pour un périmètre plus large de sociétés, par l'article 17 de la loi Sapin II. Toutefois, si la finalité préventive de ces deux dispositifs est comparable, je déplore le manque de cohérence entre eux, notamment sur le périmètre et les outils juridiques. En outre, certaines imprécisions subsistent à l'article 1. Je pense, par exemple, au champ exact des sous-traitants et fournisseurs devant être pris en compte dans le plan de vigilance. Les sous-traitants et fournisseurs de la société mère sont-ils seuls visés, ou ceux des sociétés contrôlées par la société mère le sont-ils également ? on ne peut exclure un risque d'incompétence négative du législateur ou d'atteinte au principe de clarté de la loi et à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Autre exemple faisant encourir le même risque : la rédaction ne précise pas qui pourrait mettre en demeure une société de respecter son obligation de vigilance avant une saisine du juge. Dernier exemple d'imprécision : le texte énonce que « le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale ». Le plan doit-il être élaboré en association avec les parties prenantes de la société ? Si oui, lesquelles ? Ou s'agit-il simplement d'une faculté laissée à l'appréciation de la société ? Je m'interroge, au demeurant, sur la normativité de cette disposition, alors que le Conseil constitutionnel vient de rappeler son attachement au caractère normatif de la loi. Je l'avais déjà indiqué en première lecture, les imprécisions et ambiguïtés de la rédaction

D'une part, s'agissant de l'amende civile encourue par la société en cas de manquement à l'obligation d'établir, de rendre public et de mettre en oeuvre de manière effective un plan de vigilance, la rédaction précise désormais que le montant de l'amende civile est fixé par le juge afin de se prémunir d'un risque constitutionnel au regard du principe d'individualisation des peines. Pour autant, le montant manifestement disproportionné de l'amende encourue soulève un problème sérieux de constitutionnalité. Il constitue en lui-même une atteinte aux principes constitutionnels de proportionnalité et de nécessité des peines. Une sanction ayant le caractère d'une punition doit respecter les principes du droit pénal. En l'espèce, même si elle est prononcée par le juge civil à l'occasion d'un litige entre personnes privées sur l'élaboration ou le contenu du plan de vigilance, cette amende n'en revêt pas moins le caractère d'une punition. D'autre part, s'agissant du régime spécifique de responsabilité prévu par le texte en cas de dommage susceptible de résulter d'un manquement à l'obligation d'établir, de rendre public et de mettre en oeuvre de manière effective un plan de vigilance, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture aggrave le risque constitutionnel. Cette rédaction dispose que, dans les conditions prévues par le code civil, le manquement à ces obligations « engage la responsabilité de son auteur l'oblige à réparer le préjudice que l'exécution de ces obligations aurait permis d'éviter ». Une telle formulation soulève une difficulté constitutionnelle plus grande en raison de sa portée incertaine et ambiguë et de la rupture potentielle qu'elle représente avec le principe de responsabilité tel tel que l'a consacré le Conseil constitutionnel, en dénaturant le lien de causalité entre la faute et le dommage et en pouvant faire naître un régime de responsabilité du fait de la faute d'autrui. Si l'on pouvait prétendre que la rédaction antérieure se bornait à appliquer le droit commun de la responsabilité- à tort selon moi, car il était possible d'en faire une interprétation extensive en raison de son ambiguïté -, cette nouvelle rédaction va plus loin. Comme je l'ai dit en deuxième lecture, le texte peut être compris, dans son ambiguïté, comme instaurant implicitement un régime de responsabilité pour la faute d'autrui, lequel serait évidemment contraire au principe constitutionnel de responsabilité. Le texte adopté en nouvelle lecture va plus loin et heurte davantage la conception traditionnelle et constitutionnelle du principe de responsabilité en allant au-delà de la simple responsabilité pour négligence, admise par le code civil. En outre, la mise en demeure adressée à une société de remplir ses obligations en matière de plan de vigilance, si elle peut être adressée par une association, et l'engagement de l'action en responsabilité, dans la même hypothèse, pour le compte de tiers victimes d'un préjudice, semblent heurter le principe juridique traditionnel selon lequel nul ne plaide par procureur, auquel le Conseil constitutionnel a reconnu une certaine valeur, en étant très rigoureux sur les conditions permettant à une organisation d'agir en justice pour le compte d'une autre personne, exigeant notamment le consentement de celle-ci. Enfin, l'entrée en vigueur différée de ce nouveau dispositif, introduite par le Sénat en deuxième lecture, a été approuvée dans son principe par l'Assemblée nationale, selon des modalités différentes et dans une rédaction à l'interprétation délicate. l'obligation d'établir, de publier et de mettre en oeuvre un plan de vigilance, assortie des sanctions afférentes et du régime de responsabilité, s'appliquerait « à compter du rapport [ ...] portant sur le premier exercice ouvert après la publication de la présente loi », c'est-à-dire le rapport présenté à l'assemblée générale des actionnaires en 2019, lequel portera sur l'exercice 2018, premier exercice postérieur si la loi est publiée en 2017. Mais que signifie une application « à compter d'un rapport » ? Serait-ce à compter de la publication de ce rapport ? Le Sénat avait retenu cette formulation en deuxième lecture, car il avait modifié le texte en prévoyant une obligation de publication sur les risques et les mesures de vigilance destinées à les prévenir dans le rapport du conseil. Cette formulation n'est plus adaptée au texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Ainsi, outre les objections de nature économique et pratique, toujours pleinement valables, les dispositions essentielles de la présente proposition de loi demeurent affectées par de sérieux problèmes constitutionnels que nos collègues députés n'ont pas voulu prendre en compte. L'ambition généreuse qui anime les auteurs de cette proposition de loi ne saurait conduire le législateur à méconnaître les exigences du droit. Si les grandes entreprises françaises doivent évidemment veiller aux conséquences sociales et environnementales de leur activité économique, les obligations qui peuvent leur être doivent être raisonnables et proportionnées. Elles ne sauraient se substituer à des législations étrangères insuffisantes ou à des États défaillants pour protéger leur population. En tout état de cause, il est peu probable qu'une telle législation, si elle était adoptée par la France, conduise à une amélioration de la situation sociale et environnementale des pays en développement, où sont installés nombre de sous-traitants de multinationales occidentales, ou fasse évoluer la législation de ces pays. En revanche, elle ne manquerait pas de perturber profondément le tissu économique français. Puisque les députés ont voulu conserver leur approche punitive, il est vain de persister dans notre approche de conciliation en tentant d'apporter au texte des améliorations et des clarifications. égard aux graves risques constitutionnels que recèle toujours le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, je proposerai au Sénat l'adoption d'une motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité. La parole

Encore une Lorraine ! En 2011, plus de 2 400 travailleurs se sont évanouis d'épuisement du fait de leurs conditions de travail et faute d'un salaire suffisant pour se nourrir correctement dans les usines de confection au Cambodge.

la nécessité de légiférer. Aujourd'hui, la complexité des chaînes d'approvisionnement et l'impossibilité de tenir les multinationales pour responsables des agissements de leurs sous-traitants permettent ces dérives. La France aurait pu devenir un des premiers pays à combler cette faille juridique avec la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.

En effet, comme nous l'avions indiqué, la multiplication des crises environnementales ou sociales impliquant des acteurs liés par leur activité économique impose de penser de nouvelles modalités d'encadrement, de régulation du pouvoir au sein de chaînes de valeur toujours plus complexes. Trop souvent, les multinationales, en plus de ne pas se soumettre à l'impôt, refusent tout simplement d'assumer la responsabilité civile et pénale de leurs activités. Elles créent donc des filiales toujours plus nombreuses et opaques, ont recours à une cascade de sous-traitants et se cachent derrière l'autonomie de la personne juridique quand une catastrophe humaine ou environnementale survient. Remonter la chaîne des sous-traitants et des fournisseurs dans les approvisionnements, « responsabiliser » les sociétés mères, à l'abri derrière leurs montages juridiques, tel était l'objet de la proposition de loi dont nous aurions dû débattre aujourd'hui. Nous regrettons profondément entêtement » du Sénat et du rapporteur sur ces enjeux majeurs. Comment peut-on encore penser, en 2017, que faire valoir les droits humains et environnementaux est une atteinte à la compétitivité de la France ? Comment peut-on considérer que le justifie tout ? Nous comprenons d'autant moins cette position de la commission que, comme cela a déjà été souligné lors des précédentes lectures, ce texte est au service de la compétitivité des entreprises. Loin de les fragiliser, il permettra de valoriser les efforts des sociétés vertueuses appliquant déjà des procédures d'identification et de réduction des risques. Il rétablira des conditions de concurrence plus juste en sanctionnant le social et environnemental.

Le libéralisme sans règle, c'est la jungle. Contrairement à ceux qui méconnaissent le sujet, il ne s'agit pas de gérer les entreprises, mais de leur donner un moyen compétitif supplémentaire. De nombreuses entreprises ont fait le choix du mieux-disant social et environnemental, et ce texte est là pour les encourager. Cette démarche ne fera pas fuir les investisseurs. Au contraire, elle est de nature à les rassurer. cette proposition de loi constitue un pas supplémentaire dans la lutte contre les paradis fiscaux et la fraude fiscale, car elle impose plus de transparence.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, cette nouvelle lecture de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères devrait, selon toute probabilité, faire long feu, puisque le rapporteur a déposé une motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité. Il est vrai qu'à l'issue des deux premières lectures les positions des uns et des autres,

visant à mettre les grandes entreprises face à leurs responsabilités sociales et environnementales ; d'autre part, la majorité sénatoriale demeure opposée à un texte qu'elle considère comme une entrave supplémentaire à la liberté des entreprises, dans une logique jugée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 dans le monde à mettre en place un reporting extrafinancier sur les activités de leurs sous-traitants et exécutants à l'étranger afin- c'est l'objectif affiché -de prévenir des accidents liés notamment aux mauvaises conditions de travail, comme celui survenu en 2013 au Rana Plaza, au Bangladesh, et qui a suscité une indignation internationale. En cas de manquement dans la mise en oeuvre de ce plan, l'article 2 de la proposition de loi prévoit un régime de sanction avec possibilité de mise en demeure, capacité de toute personne ayant intérêt à agir à déposer un recours en justice, réparations et amende civile pouvant atteindre désormais 30 millions d'euros. C'est donc une réforme ambitieuse, au moins sur le papier. Pour mémoire, la directive européenne de 2014 n'affiche pas le même niveau d'exigence. Un doute subsiste toutefois sur l'effectivité de cette proposition de loi. Si personne ne peut contester son bien-fondé moral, je serai pour ma part un peu plus réservé sur sa portée. En l'état actuel, de nombreuses entreprises, soucieuses de leur image, ont depuis longtemps mis en place des politiques internes en matière de RSE. Pour celles-ci, l'instauration du plan de vigilance n'apportera pas de changement majeur, si ce n'est de standardiser des pratiques qui peuvent être diverses en fonction de chaque entreprise. ce qui concerne les autres entreprises, la proposition de loi apportera une nouveauté, qui sera plus ou moins bien accueillie en fonction des ressources humaines et matérielles qui pourront être mobilisées en interne pour se mettre en conformité avec la loi. Rappelons qu'en France la jurisprudence reconnaît la compétence des juridictions françaises à juger des faits survenus en dehors du territoire français et sanctionne la négligence de la société mère de ses filiales. Des catastrophes comme l'effondrement du Rana Plaza en avril 2013 ou des pratiques moins visibles, mais malheureusement plus courantes, comme le travail des enfants, le travail des enfants, la pollution de l'environnement et, plus largement, les pratiques qui bafouent les droits élémentaires des travailleurs, devraient donc en principe être déjà condamnables en justice. Le talon d'Achille de ce texte, semble-t-il, est la territorialité du droit applicable. Car nous légiférons naturellement en droit français, pour des personnes morales

lorsqu'ils appliquent des sanctions, parfois importantes, contre des entreprises étrangères, notamment européennes, implantées sur leur sol, mais pour des activités réalisées ailleurs dans le monde. On le voit, la mondialisation, depuis une quarantaine d'années, a profondément bouleversé la notion de territoire. Les droits nationaux, européen et international s'entremêlent, en même temps que prolifèrent des zones de non-droit. Face à cette complexité inouïe, la présente proposition de loi paraît somme toute modeste. Si je ne peux que souscrire à l'intention originelle

Je regrette, à titre personnel, que l'Assemblée nationale n'ait pas choisi de rebondir sur la version adoptée par le Sénat en deuxième lecture. En restant figés sur leur texte, en ignorant les propositions du Sénat, nos collègues députés ont exclu d'avoir un débat démocratique et constructif. Pourtant, en deuxième lecture, la majorité sénatoriale avait opté pour une approche plus consensuelle visant à transposer la directive européenne d'octobre 2014.

le recours de toute personne intéressée devant le TGI en cas de manquement à ces obligations. Tous les éléments essentiels du texte étaient donc repris. Certes, nous avions supprimé l'amende civile et le régime spécifique de responsabilité, jugés excessifs et portant atteinte aux principes constitutionnels de proportionnalité et de nécessité des peines. La rédaction retenue par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture ignore ces propositions et leur visée européenne. Elle aggrave encore le risque constitutionnel. En effet, en matière de responsabilité, alors que la rédaction antérieure précisait que le non-respect des obligations concernant le plan de vigilance « engageait la responsabilité de son auteur »

Cette formulation nouvelle soulève une difficulté constitutionnelle plus grande, en raison de sa portée incertaine et ambiguë. Elle revient à dénaturer le lien de causalité entre la faute et le dommage,

adapter les modalités de la directive aux réalités des entreprises françaises, que nous voulons exemplaires, en évitant de les pénaliser excessivement et de créer des handicaps concurrentiels supplémentaires sur le marché international, tout en maintenant un objectif de vigilance. Malheureusement, cette vision responsable et pragmatique n'a pas trouvé l'écho qu'elle méritait auprès de l'Assemblée nationale, qui s'est arc-boutée sur un traitement partisan du dossier, quitte à faire peser sur les entreprises françaises des contraintes supplémentaires non seulement excessives, mais aussi exclusives. Le groupe UDI-UC adhère à l'objectif de vigilance porté par la directive européenne, mais s'oppose, vous l'avez compris, aux mesures excessives et

Monsieur le rapporteur, je veux saluer votre opiniâtreté. Après un départ en fanfare avec une motion préjudicielle, heureusement retirée, puis la suppression de tous les articles en première lecture,

Nous avions eu une petite lueur d'espoir en deuxième lecture, lorsque vous avez abandonné cette stratégie de blocage et réécrit l'article 1 de ce texte en transposant partiellement la directive sur le reporting extrafinancier. Certes, nous étions loin du compte, mais vous reconnaissiez enfin que les grandes entreprises avaient une responsabilité plus large que celle de réaliser des profits et que leur action pouvait avoir des conséquences sur la bonne marche du monde. Las, vous revenez en troisième lecture à vos premiers penchants, une obsession de l'entrave, qui nous interroge sur les puissants intérêts que protège votre groupe. Ah là là ... Cette proposition de loi trouve pourtant ses origines dans des principes internationaux auxquels la France a souscrit, quelle que soit la couleur politique de nos gouvernements. Ces textes partent du constat que les chaînes de production, de plus en plus mondialisées, engendrent une extrême fragmentation des chaînes de décision, cloisonnent les responsabilités et organisent une forme d'impunité. pour mémoire : les principes directeurs de l'OCDE proclament que les entreprises multinationales doivent respecter les droits de l'homme et parer aux incidences négatives de leur activité la déclaration de principe de l'Organisation internationale du travail et le pacte mondial des Nations unies incitent les entreprises à promouvoir les droits de l'homme dans leur sphère d'influence. Les 31 principes de Ruggie, adoptés à l'unanimité par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies, affirment que la responsabilité d'une entreprise dépasse les conséquences de ses activités pour embrasser celles de ses partenaires économiques, confirmant ainsi le lien entre maison mère, sous-traitants et fournisseurs. Cette proposition de loi s'inscrit dans une logique de transparence et d'éthique engagée en France avec la loi de 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, sous le gouvernement Jospin,

Ce texte, enfin, accompagne et généralise un mouvement volontariste du monde des entreprises, lesquelles, ayant compris que le respect de leur responsabilité sociale et environnementale est une composante de leur compétitivité, se dotent d'outils de prévention. Vous nous dites que ce texte est punitif, stigmatisant pour nos entreprises et contraire à la compétitivité. C'est faux ! Tout d'abord,

Ce texte n'est aucunement punitif, il est incitatif et préventif. Ensuite, il tend à sécuriser les entreprises en favorisant un meilleur contrôle de la chaîne de valeur, ce qui permettra d'éviter des coûts de réparation et de dédommagement en cas d'accident. Avouez qu'il est tout de même plus intelligent de consacrer des ressources à élaborer des dispositifs de prévention que de provisionner un éventuel sinistre. Enfin, nos entreprises ont compris que la mise en oeuvre de leur responsabilité sociétale est un plus en termes de compétitivité. La majorité d'entre elles s'est engagée à instaurer de bonnes pratiques, et il est regrettable que ces bons élèves soient défavorisés au regard de concurrents moins vertueux. Chers collègues, nous ne sommes plus dans le monde de Milton Friedman, qui considérait que la responsabilité sociale de l'entreprise est de faire du profit. Les entreprises vivent et prospèrent désormais dans un environnement social dont elles tiennent compte. Avoir une bonne réputation est un argument de compétitivité. L'inverse peut coûter cher. Vous nous dites également que ce texte n'est pas sûr juridiquement.

Aussi, vous l'aurez remarqué, ce texte a été sensiblement amélioré au fur et à mesure des différentes lectures, grâce à un dialogue constructif entre la société civile, le Parlement et le Gouvernement. Je voudrais à cet égard remercier les ministres concernés de leur investissement personnel et de celui de leurs services, qui nous ont permis d'aboutir à cette ultime version. Permettez-moi, pour lever toute ambiguïté, de revenir sur quelques-unes des objections que vous formulez. Vous regrettiez le flou du champ d'application des obligations de vigilance. Il a été précisé, sur le modèle de la loi Sapin II, par une liste détaillée des mesures qui devraient nécessairement faire partie du plan de vigilance.

aux entreprises agissant dans des zones de guerre soumises au terrorisme, qui devront adapter et compléter leurs mesures de vigilance, pour prévenir toute mise en cause similaire à celle, récente, d'un grand groupe français du BTP. du doigt des incertitudes s'agissant de la définition du champ exact des fournisseurs et sous-traitants. La condition de l'existence d'une « relation commerciale établie » permet de limiter le périmètre aux « partenariats dont chacun peut raisonnablement anticiper la poursuite pour l'avenir », tels que définis par la jurisprudence. Vous contestez les modalités d'élaboration du plan en association avec les parties prenantes, au nom du principe de clarté et d'intelligibilité de la loi. C'est méconnaître ce qu'est une démarche RSE, qui implique tous les acteurs de la société, au premier rang desquels les partenaires sociaux, démarche aujourd'hui maîtrisée et partagée par toutes les entreprises s'engageant dans cette voie. Vous remettez en cause le principe de proportionnalité des peines et considérez que l'amende civile de 10 millions d'euros a le caractère d'une punition. C'est éluder ce qui est écrit. L'amende encourue en cas de manquement est désormais modulée en proportion de la gravité des faits, en considération des circonstances de leur commission et en fonction de la personnalité de son auteur. 10 millions d'euros est un montant maximum en cas de défaut de plan et en l'absence de dommage. Il est donc parfaitement cohérent qu'elle puisse être portée à un maximum de 30 millions d'euros si le risque n'a pas été pris en compte et qu'une catastrophe survient. Enfin, vous considérez que le texte méconnaît le principe de responsabilité, puisqu'il permet d'engager la responsabilité d'une société du fait de la faute d'un tiers dont le lien de causalité n'est pas clairement démontré. D'une part, l'article 2 a été complété, puisqu'il est précisé que peut être engagée la responsabilité civile d'une société dont le manquement à son obligation a eu pour conséquence la survenue d'un dommage, alors que sa satisfaction aurait permis de le prévenir. D'autre part, il est D'autre part, il est désormais prévu que la procédure de sanction ne pourra être engagée qu'à l'égard d'une société préalablement mise en demeure et n'ayant pas respecté ses obligations. Cette responsabilité pourra être recherchée par toute personne ayant un intérêt à agir, comme il est d'usage en droit des sociétés. Votre dernière objection à ce texte, c'est qu'il est de portée nationale, ce qui exposerait nos entreprises à une distorsion de concurrence. Outre ce que j'ai dit précédemment sur l'intérêt pour leur réputation qu'elles peuvent tirer d'une démarche exemplaire, l'histoire montre que toutes les avancées sociales et sociétales se sont faites par la volonté politique, par la loi qui affranchit. La France, souvent en pointe en la matière, a ouvert la voie à une généralisation des bonnes pratiques. Je le rappelais en première lecture, ce fut le cas avec l'abolition de l'esclavage, avec la protection des ouvriers face aux accidents du travail, avec l'introduction de l'obligation d'une comptabilité transparente.

Chaque fois, ces mesures se sont traduites non seulement par un plus grand respect des droits humains et une amélioration des conditions de travail des salariés, mais aussi par une amélioration des performances des sociétés. Nous ne partageons pas l'idée selon laquelle les droits des ouvriers, fussent-ils au bout du monde, entraveraient la prospérité des entreprises. Nous n'acceptons pas que des enfants travaillent, que des êtres humains soient exploités, sans protection sociale ni salaire correct. Ne pas correct. Ne pas vouloir imposer ce devoir de vigilance, c'est pénaliser les entreprises vertueuses ; c'est peser à la baisse sur nos standards nationaux en matière de protection sociale, de droits des salariés, de protection de l'environnement, de lutte contre la corruption c'est inciter aux délocalisations. C'est finalement donner une prime aux mauvaises pratiques et considérer qu'elles seraient une condition de la compétitivité, ce qui n'est ni vrai ni acceptable. L'éthique est non pas un supplément d'âme, mais la raison même de l'action économique, qui fournit des biens et services dans une société qui les souhaite mais veut qu'ils soient produits en respectant les droits de l'homme et en protégeant notre planète pour les générations futures. Ce texte n'est pas un texte politique ou idéologique, contrairement à ce que vous dites. C'est un texte humaniste, au sens universel. Il aurait dû nous rassembler, mais vous avez fait le choix de l'entraver. Oui, la France est en pointe ! Oui, nous oeuvrons pour que cette loi soit suivie d'une directive européenne ! Oui, ce texte honore notre pays et rappelle notre histoire

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, mes propos ne seront guère différents de ceux que j'ai déjà tenus à plusieurs reprises sur ce texte.

d'émotion. Or l'émotion était vive lors du drame du Rana Plaza ! Aussi noble que soit ce texte, il n'aurait pas empêché un tel drame : une réponse franco-française est totalement inadaptée, surtout quand les choses évoluent continuellement aux plans européen et international. C'est pourquoi une réponse européenne et internationale est nécessaire. C'est le cas avec les principes directeurs de l'OCDE, relayés par les points de contact nationaux, les PCN, qui aident les entreprises et leurs parties prenantes à adopter une conduite responsable dans la chaîne d'approvisionnement. Le drame du Rana Plaza avait d'ailleurs donné lieu à la saisine du PCN français. Celui-ci avait rendu son rapport dès décembre 2013. 2013. Il comprenait des recommandations et des propositions pour faire évoluer les pratiques des entreprises françaises, sur la base d'un dialogue et d'un consensus entre les différentes parties : syndicat, administration, entreprise. le secrétaire d'État, pourquoi la France ne transpose-t-elle pas la directive européenne du 22 octobre 2014 relative à la publication d'informations extrafinancières ?

dans un ou plusieurs des domaines visés- informations environnementales, sociales, de personnel, de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption -devront s'en justifier publiquement. C'est là un mécanisme à la fois responsable et incitatif.

concurrentielle. Une réponse franco-française à la question posée n'est pas adaptée. C'est bien là l'erreur majeure du présent texte ! Je rappelle d'ailleurs que les entreprises françaises ont d'excellents résultats en matière de RSE, Une étude du mois de mars 2015, menée par EcoVadis et la médiation interentreprises, montre que la France fait figure de leader mondial en la matière

La situation de l'emploi est-elle si florissante ? Les entreprises françaises sont-elles en si bonne santé ?

faible, mais ces 243 entreprises représentent en réalité plus de 4 millions de salariés, plus de 33 % de la valeur ajoutée produite en France et plus de 50 % du chiffre d'affaires à l'export ! Il est donc aisé de comprendre que la proposition de loi aurait un effet sur de très larges pans de l'économie française. En outre, sur le plan pratique, les entreprises seraient confrontées à l'impossibilité de mettre en oeuvre cette obligation de vigilance sur toute leur chaîne de sous-traitants et de fournisseurs. Telle est la réalité, en particulier, pour les TPE et PME françaises.

de l'entreprise, qui n'aurait pas été en mesure de le prévenir. Or les entreprises françaises ne cessent d'attirer notre attention sur le poids du fardeau administratif, qu'elles nous demandent avec insistance d'alléger. Par ailleurs, les fragilités juridiques du texte sont nombreuses. Nous les avons soulignées au fil des débats. Nous avons également mis en exergue les principes constitutionnels que cette proposition Quoi qu'il en soit, le groupe Les Républicains du Sénat ne peut soutenir un texte qui promeut une vision idéologique de l'entreprise. Évitons la caricature d'un chef d'entreprise irresponsable et irrespectueux du droit de la protection des salariés et de l'environnement

Aucune entreprise n'a les moyens de savoir ni ce que doit comporter le plan de vigilance ni quelles sont les mesures de « vigilance raisonnable » qui doivent être mises en oeuvre. Le renvoi à un décret ne règle pas cette question

L'article 34 de la Constitution dispose que la loi détermine les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale tombe sous le coup du grief d'incompétence né de l'article 34 de la Constitution. En outre, la proposition de loi viole les exigences constitutionnelles applicables en matière de sanctions : le Conseil constitutionnel a rappelé à plusieurs reprises que le principe de légalité des délits et des peines s'applique aux amendes civiles lorsqu'elles ont la nature de sanctions ayant le caractère d'une punition. Il a décidé que les principes découlant des articles VIII et IX de la Déclaration de 1789 sont applicables à ces amendes. L'amende civile prévue par le texte de l'Assemblée nationale, laquelle peut aller jusqu'à 10 millions d'euros, constitue une sanction ; elle doit donc respecter le principe de légalité pénale. implique un impératif de précision, que le texte ne respecte pas, ni en matière de définition du champ d'application ni en matière de qualification juridique de l'infraction et du référentiel applicable. De la même façon, le texte ignore le principe constitutionnel d'égalité. En effet, seules les entreprises dont le siège est domicilié en France seront affectées par ce texte. Celles de leurs concurrentes dont les sièges sociaux sont établis hors de France pourront continuer à vendre sur le territoire français des produits ne répondant pas aux mêmes exigences. Enfin, la proposition de loi se heurte à la garantie des droits. Lorsqu'un dommage surviendra du fait d'une filiale ou d'un sous-traitant, les sociétés mères seront considérées comme coupables de ne pas avoir conçu ou mis en oeuvre un plan de vigilance suffisant. Mais elles ne disposeront d'aucune possibilité de dégager leur responsabilité en démontrant leur absence d'implication ou de faute. Je ne développerai pas davantage mon propos ; mon collègue Christophe-André Frassa l'a très bien fait. Vous l'aurez compris : le groupe Les Républicains votera pour la motion.

Les arguments que vous avez donnés, madame la vice-présidente de la commission des lois, ne nous paraissent absolument pas pertinents.

Monsieur Guillaume, vous y avez siégé ! « Pour les propositions de loi sénatoriales inscrites en première lecture dans les espaces réservés et sauf accord du groupe auteur de la demande d'inscription La commission ne peut modifier le texte de la proposition de loi (et, à défaut, elle ne peut que le rejeter pour permettre son examen article par article en séance publique). « La commission et les sénateurs s'abstiennent de déposer l'exception d'irrecevabilité même si, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, doit être préservée la possibilité effective, pour les parlementaires, de contester la conformité à la Constitution des dispositions d'un texte ; « la question préalable la motion de renvoi en commission ou la motion préjudicielle, qui ont pour effet de suspendre la navette et pourraient être considérées comme contradictoires avec le droit des groupes à voir discuter en séance les sujets qu'ils proposent dans leur espace réservé. Pour permettre le débat en séance publique, le texte est examiné article par article. « Pour tous les autres textes inscrits dans les espaces réservés : « Commissions et sénateurs peuvent exercer la plénitude de leur droit d'amendement. Exception d'irrecevabilité et question préalable sont recevables à chaque stade de la procédure. Elles peuvent être discutées après la discussion générale si le groupe auteur de la demande d'inscription le souhaite. La commission et les sénateurs s'abstiennent, sauf accord du groupe auteur de la demande d'inscription, de déposer la motion de renvoi en commission ou la motion préjudicielle, qui ont pour effet de suspendre la navette et pourraient être considérées comme contradictoires avec le droit des groupes à voir discuter en séance les sujets qu'ils proposent dans leur espace réservé.

Le scrutin est clos.

prises pour son application, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a émis un avis défavorable- 10 voix pour, 16 voix contre, 2 bulletins blancs -à la nomination de M. Philippe Martin aux fonctions de président du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables renouvelables est parvenue à un texte commun. L'ordre du jour appelle la discussion, à la demande du groupe du RDSE, de la proposition de loi visant à mettre en place une stratégie nationale d'utilisation du transport sanitaire héliporté

On pense d'emblée, bien sûr, aux territoires ruraux ou aux territoires de montagne. Mais ce texte concerne aussi la ville. Interrogé sur le sujet en 2012, l'éminent géographe Emmanuel Vigneron

des territoires : les Ardennes, la Moselle, le Doubs, la Haute-Savoie, la Savoie, les Alpes-Maritimes, les deux départements de la Corse, les Landes, la Loire-Atlantique, les Pyrénées-Orientales, la Lozère et même, tout près de Paris, l'Oise et la Seine-Maritime.

Troendlé sur l'évolution de l'activité des services départementaux d'incendie et de secours en matière de secours à personne, datant du mois d'octobre 2016. Selon ces collègues, « la politique d'emploi des hélicoptères n'est ni claire ni logique.

Pierre-Yves Collombat et Catherine Troendlé remarquaient dans leur rapport qu'« une part de l'activité du groupement des hélicoptères de la sécurité civile relève de la décision des seuls SAMU, sans aucun droit de regard sur le bien-fondé de leur demande.

dans un service unifié placé sous l'autorité du Premier ministre. Je n'oublie pas non plus le rapport du Conseil national de l'urgence hospitalière qui a dressé une liste de recommandations visant à obtenir un maillage territorial uniforme. Les auteurs de ce document demandaient une véritable stratégie nationale prévoyant une organisation, un schéma et un type de fonctionnement adapté dans chaque région, et qui serait partagée par l'ensemble des acteurs du transport sanitaire héliporté. Tout cela est de bon sens. Fort de l'appui de ces deux rapports pertinents, précieux et circonstanciés, je

De manière un peu poétique, mais aussi très pratique, le professeur Pierre Carli, médecin-chef du SAMU de Paris, m'a confié lors de son audition que chaque hélicoptère du SAMU avait son histoire.

Ce sont donc les collectivités territoriales- les villes, les départements, les régions -, parfois plusieurs d'entre elles, parfois une seule, car un maire ou un président est particulièrement impliqué, qui permettent de mettre en place le financement nécessaire pour que l'équipe d'urgence dispose de moyens héliportés. Cela a été dit, en France, à l'heure actuelle, 45 hélicoptères sont affectés aux SAMU. pour deux types de missions. Les missions dites de soins primaires, d'abord, qui impliquent de se rendre sur le lieu de la prise en charge des personnes malades ou blessées pour assurer le transport de celles-ci vers les services d'urgence. Les missions dites secondaires, ou plus exactement de second temps, ensuite, à savoir le transport des patients entre hôpitaux pour permettre la prise en charge la plus adéquate. Ces transports secondaires ne sont pas nécessairement urgents ; ils peuvent être programmés. La distinction entre ces deux missions doit être relativisée, car certains patients sont d'abord dirigés vers l'hôpital le plus proche pour y être stabilisés, diagnostiqués, avant d'être éventuellement orientés par hélicoptère, en fonction de l'urgence, vers l'établissement disposant du plateau technique adapté à leur état.

et par là même renforce le besoin en moyens de transport médicalisés et rapides. L'attractivité de l'hélicoptère est donc forte. Les moyens en hélicoptères sont cependant mal répartis et le mode de financement des Héli-SMUR rend la gestion de ces derniers complexe. Les appareils sont loués à des entreprises qui assurent l'entretien technique et emploient les pilotes. Les possibilités techniques de ces appareils ainsi que le niveau d'habilitation des pilotes restreignent souvent l'usage qui peut en être fait. Les médecins régulateurs des SAMU, les seuls à pouvoir décider d'une intervention médicale d'urgence, ont donc régulièrement recours aux autres hélicoptères de secours disponibles, essentiellement ceux de la sécurité civile. Les hélicoptères de la Les hélicoptères de la gendarmerie n'interviennent en effet pour les secours à personne que dans le cadre historiquement délimité du secours en haute montagne. La question qui se pose est donc essentiellement celle de l'articulation entre les Héli-SMUR et les hélicoptères de la sécurité civile. On estime effectivement que près de la moitié des hélicoptères de la sécurité civile sont en pratique employés pour des activités de transport sanitaire. Ce sont des appareils plus polyvalents, dont les pilotes sont hautement entraînés et habilités notamment au vol de nuit, ce qui n'est pas le cas des Héli-SMUR. Si le SAMU peut faire appel aux hélicoptères de la sécurité civile, il ne peut cependant en disposer à sa guise. Les appareils ne sont pas forcément basés à proximité des hôpitaux. Surtout, ils sont prioritairement affectés aux missions de sécurité civile pour lesquelles ils ont été créés, et ne sont donc pas toujours disponibles. Logiquement, du côté tant des SMUR que de la sécurité civile,

C'est aussi l'objet de la proposition de loi déposée par Alain Bertrand, Jacques Mézard et les membres du groupe du RDSE, dont nous sommes saisis aujourd'hui. La commission des affaires sociales a estimé que ce texte posait une vraie question et appelait une réponse du législateur. Elle a cependant considéré qu'il était nécessaire de se garder de plusieurs risques. En effet, il ne faut pas céder à la tentation d'un « hélicentrisme » exagéré. Tous les acteurs en sont d'accord, l'hélicoptère n'est qu'un moyen parmi d'autres pour le transport sanitaire et, même dans les cas d'urgence, il n'est pas toujours le plus approprié. Accessoirement, il est relativement coûteux. Entre le moment où le médecin régulateur des urgences reçoit l'appel et celui où l'hélicoptère peut arriver sur les lieux, plusieurs retards peuvent se cumuler.

Par rapport aux véhicules terrestres, l'avantage n'est donc pas toujours établi. De nuit, quand les routes sont dégagées, le transport par un véhicule du SMUR peut aller plus vite que le transport par un hélicoptère pas forcément disponible immédiatement. Il faut donc utiliser l'hélicoptère quand il présente un avantage évident. On ne peut l'envisager indépendamment des transports sanitaires terrestres. Inversement, si l'engagement pris de permettre partout sur le territoire l'accès aux soins urgents en moins d'une demi-heure fait sens en termes sanitaires, il n'est pas pertinent pour tous les déplacements programmés entre hôpitaux. Comment parvenir Comment parvenir à la gestion optimale des moyens héliportés ? aboutissait de fait à transférer une part importante des hélicoptères de la sécurité civile aux SAMU. Cette solution avait certes le mérite de la cohérence sur le plan sanitaire, mais elle a paru à la commission difficilement applicable sur le terrain. la commission a adopté, sur mon initiative, un amendement tendant à reprendre la solution préconisée par Catherine Troendlé et Pierre-Yves Collombat dans leur rapport. Il s'agit de prévoir la mutualisation de tous les hélicoptères par un service rattaché au Premier ministre, un service ne dépendant donc ni du ministère de l'intérieur ni de celui de la santé. Très bien ! Ce service serait chargé de l'implantation des appareils. La gestion de ceux-ci serait faite à l'échelon le plus adéquat, peut-être la région. Les objectifs assignés à ce service seraient ainsi d'assurer le maillage territorial et de garantir l'accès aux urgences en moins de trente minutes. Il me semble que cette mesure, qui n'entrave pas les solutions déjà trouvées sur le terrain et ne préjuge pas du mode de gestion territorial le plus adéquat, peut être un point d'équilibre. La parole est à Mme

Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui aborde une question essentiellement opérationnelle l'aide médicale urgente réalisée par Héli-SMUR et les interventions réalisées par les hélicoptères d'État de la sécurité civile, notamment dans le cadre du secours à personne. Elle a pour objet de demander la mise en place d'une gestion mutualisée de ces deux flottes d'appareils. En ce qu'ils contribuent à garantir l'accès aux soins urgents de la population en moins de trente minutes, comme s'y était engagé le Président de la République en 2012, les hélicoptères d'État et les hélicoptères des établissements de santé représentent un enjeu majeur pour l'accès aux soins urgents sur le territoire national. Il est en effet nécessaire d'optimiser l'utilisation du vecteur héliporté, afin d'améliorer la complémentarité, la cohérence et l'efficacité du recours aux différentes flottes.

toutes choses, je souhaite rappeler que le secours à personne et l'aide médicale urgente recouvrent des champs distincts, mais complémentaires. L'aide médicale urgente et le secours à personne sont en effet des missions de service public différentes par leur objet ; néanmoins, elles se complètent dans leur finalité : le service des mêmes usagers, patients ou victimes. L'aide médicale urgente, mission de service public hospitalier, a pour objet d'assurer aux malades, blessés ou parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état. Le secours à personne, quant à lui, est l'une des missions de sécurité civile assurée principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services départementaux d'incendie et de secours. Il vise notamment à assurer la mise en sécurité des victimes, à pratiquer les gestes de secourisme en équipe et à réaliser l'évacuation éventuelle de la victime vers un lieu d'accueil approprié. Si les Héli-SMUR sont entièrement dédiés à l'aide médicale urgente, les missions remplies par les hélicoptères de la sécurité civile ne se bornent pas aux missions de secours à personne et d'aide médicale urgente. Elles englobent le champ plus vaste de la protection des personnes et des biens, avec des missions complémentaires telles que la lutte contre les feux de forêt, la projection d'équipes spécialisées, ou la participation à des missions de sécurité publique. La structure de commandement de ces moyens et leur cartographie d'implantation découlent d'ailleurs de cette pluralité de missions. Je l'ai dit en introduction, nous partageons largement l'objectif de complémentarité des moyens héliportés ; c'est le sens du travail interministériel déjà engagé. Si l'aide médicale urgente relève de la compétence du ministère de la santé, et si les missions de sécurité civile relèvent de celle du ministère de l'intérieur, la coordination des interventions, la complémentarité des moyens et, plus généralement, la coopération des services constituent un impératif. Cette coopération se réalise déjà au quotidien, à travers, notamment, la participation quotidienne des hélicoptères de la sécurité civile aux missions d'aide médicale urgente. Il est toutefois possible d'aller plus loin. Le travail interministériel qui a déjà été engagé sur les Héli-SMUR et les hélicoptères de la sécurité civile traduit la volonté de renforcer la complémentarité de ces moyens. En effet, l'axe 2 de la feuille de route santé-intérieur de 2014 a fixé comme objectif de « renforcer les outils permettant d'assurer la complémentarité des moyens humains et matériels, tant terrestres qu'héliportés. Dans cette optique, un comité de pilotage interministériel dédié précisément à la complémentarité des moyens héliportés utilisés dans le cadre du secours à personne et de l'aide médicale urgente a été mis en place. La direction générale de l'offre de soins, la DGOS, et la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, la DGSCGC, finalisent actuellement une instruction interministérielle relative à la complémentarité des Héli-SMUR et des hélicoptères d'État. Ce document identifiera des principes partagés de complémentarité, de cohérence, d'efficience, de transparence, ainsi que des indicateurs communs d'activité des moyens héliportés. détaillera également les modalités d'implantation et de fonctionnement des bases, ainsi que les principes de mise en oeuvre opérationnelle des moyens, c'est-à-dire, concrètement, l'emploi de l'hélicoptère le plus adapté à la mission et disponible dans les délais compatibles avec l'état du patient. Enfin, cette instruction interministérielle posera les principes de gouvernance à l'échelon national comme territorial. Mais, sur le terrain, les avancées sont d'ores et déjà notables dans plusieurs régions, avec un engagement fort des directeurs généraux des agences régionales de santé et des préfets, dans la droite ligne de la feuille de route santé-intérieur.

l'articulation des deux flottes Héli-SMUR et sécurité civile est déjà active pour la période nocturne, ce qui permet la couverture d'anciennes zones blanches. Pour aller encore plus loin sur ce sujet, le Gouvernement a également souhaité qu'une revue des dépenses soit conduite au mois de mai 2016 sur le thème des hélicoptères de service public, par une mission inter-inspections réunissant l'Inspection générale des finances, l'Inspection générale de l'administration, l'Inspection générale des affaires sociales et le contrôleur général des armées. La mission a salué le travail interministériel conduit par les ministères de la santé et de l'intérieur pour améliorer la cohérence d'emploi des hélicoptères, ainsi que la complémentarité de l'utilisation des moyens. Si les recommandations de la mission font actuellement font actuellement l'objet d'une réflexion approfondie et partagée entre les administrations, il est intéressant de relever qu'elles comprennent non pas la mutualisation des flottes, mais l'amélioration de la coordination des moyens. J'en viens maintenant au contenu de la proposition de loi que nous examinons. Tout d'abord, je tiens à saluer la cohérence de la commission des affaires sociales, dont le Gouvernement souscrit pleinement à l'analyse concernant le contenu

En réécrivant l'article unique de ce texte, la commission des affaires sociales, par la voix de son rapporteur, a proposé la création d'un service placé auprès du Premier ministre, service qui serait chargé de la gestion mutualisée des hélicoptères.

pour renforcer la cohérence et l'efficience du système. C'est la direction préconisée par les travaux menés conjointement par la DGOS et par la DGSCGC, et sur lesquels la revue de dépenses s'est en partie fondée. Par ailleurs, vous avez vous-même soulevé lors de l'examen en commission le risque d'« hélicentrisme », puisque la proposition de loi que nous examinons semble inciter à faire reposer l'accès aux soins d'urgence prioritairement sur le vecteur héliporté, sans aborder la complémentarité avec les autres vecteurs terrestres maritimes. Actuellement, si l'accès aux soins urgents en moins de trente minutes est assuré pour quasiment 100 % de la population- 98,5 % exactement -, c'est parce que nous prenons en compte l'ensemble des services d'urgence, SMUR, médecins correspondants du SAMU, Héli-SMUR et hélicoptères de la sécurité civile. Ce résultat montre bien que les hélicoptères sont des vecteurs complémentaires des vecteurs de l'aide médicale urgente. Il ne faut pas oublier que ces derniers ont leurs propres contraintes, notamment le respect des conditions minimales de vol et de la réglementation aérienne. que le texte que nous examinons, en prévoyant une gestion mutualisée des Héli-SMUR et des hélicoptères de la sécurité civile sous l'angle unique de l'accès aux soins d'urgence, apporte une réponse incomplète à la problématique globale des hélicoptères de service public. En effet, les hélicoptères de la sécurité civile ne sont pas les seuls hélicoptères d'État à participer aux missions de secours à personne et d'aide médicale urgente. C'est aussi le cas d'une partie de la flotte de la gendarmerie nationale, notamment en zone de montagne et en outre-mer, mais aussi d'une partie de la flotte de la marine nationale et de l'armée de l'air. Ces flottes ont en commun d'avoir des missions qui ne sont pas limitées au secours à personne et à l'aide médicale urgente. Leur localisation et leurs chaînes de commandement répondent à la diversité de ces missions, dans des logiques d'articulation avec d'autres moyens qui sont propres à chaque service. une régulation de l'offre des vecteurs héliportés, telle qu'elle est inscrite dans la proposition de loi à un niveau central, serait en décalage avec les missions déléguées aux ARS dans l'organisation et la régulation de l'offre de soins, je pense en particulier à l'attribution et au renouvellement des autorisations d'activité des structures d'urgence. Le principe de subsidiarité en faveur des représentants de l'État en région- les préfets et les directeurs généraux des ARS -doit prévaloir avec l'appui de chaque ministère. Mesdames, messieurs les sénateurs, le travail de coordination que vous appelez de vos voeux avance et va se poursuivre, avec la publication prochaine de l'instruction interministérielle que j'ai annoncée. annoncée. Si le Gouvernement partage la volonté de mieux coordonner encore les moyens aériens pour mieux couvrir nos territoires, les outils législatifs ou réglementaires qui seraient nécessaires ne peuvent précéder la fin des travaux actuellement menés entre les acteurs opérationnels. Vous l'aurez donc compris, le Gouvernement n'est pas favorable à l'adoption de cette proposition de loi qui pourrait compromettre l'ensemble des travaux engagés par le ministère de la santé

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la proposition de loi initiale présentée par les membres du groupe du RDSE visait à améliorer les transports sanitaires héliportés en mettant en place une instance régionale, la commission régionale des transports héliportés, chargée d'établir un schéma d'implantation des hélicoptères avec pour objectif un accès aux soins trente minutes maximum. En effet, le transport sanitaire héliporté est parfois la solution la plus rapide pour les malades d'accéder aux soins urgents dans nos territoires ruraux et de montagne. Lorsque l'hôpital le plus proche se situe au-delà d'une heure de trajet, seul l'hélicoptère permet une évacuation rapide des personnes malades ou blessées. Or, on le sait bien, les chances de survie du patient ou la gravité des séquelles sont strictement corrélées au temps de transfert. Il est donc nécessaire de prévoir une prise en charge la plus rapide possible.

en moins d'une demi-heure. Ainsi, la proposition de loi initiale prévoyait de mettre en place une stratégie nationale d'utilisation du transport sanitaire héliporté, déclinée à l'échelon régional par des contrats de mission santé entre l'État et les prestataires, afin de garantir afin de garantir une prise en charge en trente minutes. L'objectif étant d'optimiser les moyens et l'implantation des transports sanitaires héliportés pour améliorer le fonctionnement et la qualité de soins, cette organisation était censée être pilotée par l'ARS grâce à la création d'une commission régionale des transports

Néanmoins, en commission, le rapporteur, Gilbert Barbier, lui aussi membre du groupe du RDSE, a complètement réécrit cette proposition de loi. La nouvelle rédaction convient à Alain Bertrand et aux membres de son groupe. C'est donc de cette nouvelle version que nous allons débattre. prévoit désormais que la gestion des hélicoptères pour le transport sanitaire d'urgence sera mutualisée et sera réalisée à l'échelon national, par un service placé auprès du Premier ministre.

collègues, au travers de cette proposition de loi, c'est bien la question de l'accès aux soins d'urgence qui est posée et non pas seulement celle d'une meilleure organisation des transports sanitaires héliportés. De fait, une meilleure De fait, une meilleure articulation entre les Héli-SMUR et les hélicoptères de la sécurité civile constitue un remède aux économies réalisées sur la santé et la sécurité sociale. Avec la réduction de l'offre de soins, les fermetures des établissements de santé et les groupements hospitaliers de territoire, les GHT, la distance entre les habitants et les hôpitaux s'est allongée au détriment de la bonne santé des individus.

Aussi, loin de régler la problématique des déserts médicaux, ces GHT vont accentuer les inégalités en matière de densité médicale et paramédicale dans les régions ». Cela risque, par conséquent, d'accentuer les inégalités d'accès aux services d'urgence.

Au contraire, les collectivités territoriales, qui subissent le désengagement financier de l'État, doivent toujours se débrouiller seules pour trouver les fonds nécessaires à l'acquisition et à la maintenance des flottes aériennes. En conclusion, malgré ces critiques sur les limites de ce texte, qui tend à améliorer l'organisation du transport héliporté, mais ne remet pas en question le désinvestissement de l'État dans le financement de nos hôpitaux, nous voterons en faveur

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le transport sanitaire héliporté fait partie de notre système de soins d'urgence. Il est indéniable qu'il permet de par sa rapidité une amélioration de la qualité et de la sécurité des soins d'urgence. Deux typologies de transport doivent être distinguées : le transport primaire, qui permet l'évacuation d'un accidenté ou d'une victime vers un lieu de prise en charge adapté ; le transport secondaire, qui permet d'assurer dans les plus brefs délais le transfert d'un patient d'un établissement vers un autre. Deux organisations de moyens héliportés cohabitent également dans notre dispositif de secours et d'intervention. L'une basée sur l'utilisation d'hélicoptères privés mis à disposition et adaptés aux missions des équipes des SAMU et des SMUR : les Héli-SMUR. L'autre fondée sur l'utilisation d'hélicoptères d'État, agencée autour de la notion de secours à personne, et gérée par la sécurité civile. Chaque système comporte des avantages et des inconvénients. les Héli-SMUR, la disponibilité des appareils étant permanente, l'équipe SMUR n'étant mobilisée que pour la durée de la mission, elle peut participer à d'autres tâches hospitalières ; le matériel médical, quant à lui, est à poste fixe dans l'hélicoptère, ce qui réduit les délais de préparation. L'Héli-SMUR s'adapte parfaitement au fonctionnement du système de soins. En revanche, son statut privé lui impose de se conformer strictement à la réglementation aérienne civile. Le type d'appareil utilisé par Héli-SMUR ne permet pas de missions en milieu périlleux ou en cas de visibilité diminuée. Concernant les hélicoptères d'État, leur principal avantage réside dans leur statut dérogatoire et leur potentiel. Des inconvénients doivent cependant aussi être évoqués. Tout d'abord, l'exercice non exclusif et non prioritaire de la mission sanitaire est un réel problème. En effet, les hélicoptères sont partagés entre sécurité civile, gendarmerie, marine nationale et armée de l'air, et sont placés sous contrôle du préfet de la zone de défense. Aussi, leur positionnement a été réalisé pour répondre à ces diverses missions. l'entourage technique et l'absence de régulation médicale compliquent leur utilisation. Enfin, leur financement est totalement pris en charge par le ministère d'origine ; cette apparente gratuité ne permet pas d'afficher le coût réel des interventions sanitaires et donc de budgéter leur financement. Cependant le coût d'un hélicoptère de la sécurité civile est évalué à environ 3 500 euros par heure de vol, hors coût de l'équipe médicale. L'exercice qui nous est proposé aujourd'hui par nos collègues du groupe du RDSE porte sur la pertinence et sur l'optimisation des moyens. en évidence les auteurs de cette proposition de loi, il n'existe actuellement aucune stratégie nationale clairement définie. C'est cette absence de stratégie nationale qui explique les disparités régionales d'implantation des Héli-SMUR, mais également l'absence de complémentarité avec les hélicoptères de la sécurité civile. À ce jour, l'implantation des appareils n'est pas optimisée ; elle est même insuffisante dans certaines régions. Nos collègues, auteurs de la présente proposition de loi, partent du constat que dans de nombreux territoires, souvent ruraux et de montagne, mais pas seulement, peu d'hôpitaux et de maternités sont en mesure d'offrir tous les types de soins appropriés à toutes les urgences. Il faut donc transférer les patients dans des hôpitaux plus grands. Dans ces conditions, les transferts sanitaires peuvent être très longs, et durer entre une heure et une heure trente. Le transport héliporté se pose alors en alternative, ce moyen permettant de relier le grand hôpital le plus proche en moins de trente minutes. L'amélioration du système actuel impose une évolution de l'organisation et de la réglementation. L'article unique de cette proposition de loi vise à créer notamment à l'échelon national un contrat de mission santé élaboré par l'État, et qui s'imposera à l'ensemble des prestataires et des intervenants dans le cadre du transport sanitaire héliporté, donnant ainsi priorité à la mission sanitaire. Le Conseil national de l'urgence hospitalière énumère parfaitement les principaux points du contrat de mission santé l'hélicoptère de la mission santé est dédié spécifiquement à cette tâche et à un positionnement hospitalier ; de plus, la régulation médicale des transports sanitaires est effectuée par le SAMU ; ensuite, la médicalisation de l'hélicoptère sanitaire est assurée par une équipe SMUR ou garantissant le même niveau de soins enfin, l'équipe SMUR est à tout moment disponible pour médicaliser l'hélicoptère, mais elle n'est pas exclusivement dédiée à cette tâche pour garantir l'efficience de l'usage du temps médical. Par ailleurs, confier aux agences régionales de santé l'organisation du transport sanitaire à l'échelon régional devrait avoir pour objectif de garantir l'essentiel du contrat de mission. Il semble indispensable de regrouper acteurs et utilisateurs à l'échelle territoriale. Les ARS devront par conséquent entreprendre un programme de recensement, d'amélioration et, si nécessaire, de création de zones à poser. Elles pourront établir une cartographie précise de la couverture optimale de la région et un schéma d'implantation des hélicoptères répondant mieux aux besoins des différents territoires en termes de population, d'infrastructures, de risques particuliers, ou encore de saisonnalité des besoins.

Ce coût est inférieur à celui d'un hélicoptère de la sécurité civile avec une moyenne de 1,75 million d'euros par an hors coût de l'équipe médicale. Concernant les Héli-SMUR, le budget régional consacré aux hélicoptères est très variable d'une région à une autre, allant de 300 000 euros à plus de 8 millions d'euros. Aussi, nous devons travailler à la pérennisation et à l'uniformisation du financement des hélicoptères sanitaires. Le constat partagé que nous faisons, mes chers collègues, porte sur l'utilisation des hélicoptères sanitaires et sur l'existence de disparités importantes en matière de couverture du territoire, les modalités d'utilisation de l'hélicoptère étant tributaires de son statut et non de sa mission sanitaire ! Cette nouvelle organisation nécessitera une adaptation des services existants très bien définie par le Conseil national de l'urgence hospitalière. pour les hélicoptères d'État, le contrat mission santé va impliquer un effort en termes d'organisation et de répartition des moyens héliportés. La mission sanitaire, jusque-là complémentaire, deviendrait une mission principale pour ces hélicoptères, qui seraient intégrés dans le dispositif des transports sanitaires héliportés. Le repositionnement des hélicoptères d'État et des infrastructures nécessaires devra donc être envisagé pour améliorer la couverture de certaines régions, et ainsi pour qu'ils soient complémentaires des moyens existants. pour les Héli-SMUR, la dimension régionale, la mutualisation et la transparence des missions doivent être développées ou améliorées. Les prestations de services, quant à elles, doivent être standardisées. Une stratégie nationale de couverture du territoire est essentielle et elle doit passer par deux axes : remettre le patient au centre du système, avec la mise en place du contrat de mission santé ; confier aux ARS l'organisation des transports sanitaires héliportés comme pour tout dispositif de soins. Cela se traduit, bien sûr, par une organisation régionale partagée par différents acteurs et intervenants. Je veux saluer la clairvoyance et l'initiative tout à fait intéressante du rapporteur, Gilbert Barbier,

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'accès aux services sanitaires, en particulier hospitaliers d'urgence, est certes une réalité pour les habitants des grandes agglomérations, dont je suis un représentant, mais elle demeure une attente très mal satisfaite pour les autres. Cette disparité profonde ne date pas d'aujourd'hui. Elle a pris forme dès 1958 avec la création des centres hospitaliers et universitaires.

des premiers schémas régionaux d'organisation sanitaire à partir de 1994. Je ne veux pas entrer dans le débat de savoir s'il était utile ou pas de regrouper des établissements hospitaliers et de rationaliser le nombre de lits d'hospitalisation, afin de réaliser des économies d'échelle.

que soit intégré dans ce calcul le coût d'acheminement rapide des accidentés graves et des grands malades vers les centres hospitaliers compétents. Il faut un personnel médical extrêmement qualifié et disponible, il faut aussi un outillage médical et chirurgical de pointe. Ces exigences peuvent en partie justifier le fait d'avoir opéré certains regroupements de structures hospitalières. C'est parfois aussi l'argument qui est avancé pour légitimer une logique purement comptable au détriment de l'égalité de chacun face à la souffrance, de l'égalité des territoires et de l'égalité de traitement qui doit fonder l'existence d'un service public. En effet, la contrepartie bien visible de ce long processus de regroupement a été de créer, voire de renforcer, ces fameuses zones blanches sans lieu d'accueil médical. Face à cette inégalité flagrante de traitement, Alain Bertrand et les membres du groupe du RDSE nous proposent de rationaliser le transport sanitaire héliporté, afin de permettre à toutes les personnes en état d'urgence de bénéficier de soins. Nous ne pouvons que les remercier de cette juste initiative, ! On parle de nouveau et de plus en plus, notamment grâce au Sénat, de « déserts médicaux ». Il s'agit d'une terrible réalité qui touche bien sûr les espaces les plus ruraux et les plus montagneux de l'Hexagone.

qui, en la matière, règnent dans certains de nos départements et certaines de nos régions d'outre-mer. Un accidenté grave en Guyane a encore moins de chance de pouvoir être pris en charge qu'en France métropolitaine. J'ai bien conscience que l'usage d'un hélicoptère même rationalisé pour des raisons médicales

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons une proposition de loi de MM. Alain Bertrand et Jacques Mézard, et des membres du groupe du RDSE, visant à mettre en place une stratégie nationale d'utilisation du transport sanitaire héliporté. Je veux remercier tout d'abord Gilbert Barbier de son rapport approfondi et mesuré. L'objet de cette proposition de loi est donc de mettre en place une stratégie nationale d'utilisation du transport sanitaire héliporté. Dans la version initiale de ce texte, l'organisation en revenait aux agences régionales de santé, l'objectif étant de permettre un transfert primaire- prise en charge de patients

au sein du SAMU 62 : il dispose depuis plus de vingt-cinq ans d'un hélicoptère sanitaire, financé au départ par l'État et le conseil général du Pas-de-Calais. À ce jour, il n'existe plus que des crédits d'État déconcentrés à l'échelon de l'agence régionale de santé. Dès son implantation, cet hélicoptère a surtout concerné le transport secondaire, le Pas-de-Calais, département de 1,5 million d'habitants ne disposant pas de centre hospitalo-universitaire, mais bénéficiant de sept SMUR implantés dans ses sept hôpitaux généraux. Cela permet une bonne couverture pour le transport primaire quand, par ailleurs, les relations entre le SAMU et les sapeurs-pompiers sont excellentes. Ainsi, en 2014, cet appareil a effectué 703 heures de vol, 1 heure par mission, 75 % de transports secondaires, 25 % de transports primaires,

cet hélicoptère, loué à une société belge, répond totalement aux normes de sécurité européennes, puisqu'une personne de surveillance des fonctions techniques

Nos travaux en commission ont permis d'améliorer le texte sous l'impulsion du rapporteur, qui a proposé un amendement de réécriture globale de l'article unique de cette proposition de loi. L'article unique modifié prévoit une gestion mutualisée par un service placé auprès du Premier ministre des hélicoptères susceptibles d'assurer le transport sanitaire, afin de garantir la répartition de ceux-ci sur le territoire. La gestion des hélicoptères serait faite à l'échelon territorial le plus adapté, en coordination avec les possibilités de transports terrestres. Elle préserverait la compétence du médecin régulateur pour décider de la nécessité d'un transport héliporté, ce que nous approuvons. Cependant, Mme Bricq nous a alertés sur un point. On peut en effet s'interroger sur l'efficacité d'une délégation interministérielle placée auprès du Premier ministre d'une délégation interministérielle placée auprès du Premier ministre entre les agences régionales de santé et les préfets de département pour assurer une coordination de l'utilisation des transports héliportés.

C'est l'objectif de l'axe 2 de la feuille de route santé-intérieur de 2014, à savoir « renforcer les outils permettant d'assurer la complémentarité des moyens humains et matériels, tant terrestres qu'héliportés. La direction générale de l'offre de soins et la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ont mis en place un comité de pilotage interministériel dédié à la complémentarité des moyens héliportés utilisés dans le cadre du secours à personne et de l'aide médicale urgente, le SAP-AMU, les Héli-SMUR et les hélicoptères de la sécurité civile. Cette structure est le lieu de concertation interministérielle sur ces questions d'intérêt commun. Les deux directions viennent de s'accorder sur un texte conjoint relatif à la complémentarité des moyens héliportés qui sont utilisés dans le cadre du SAP-AMU, Héli-SMUR et hélicoptères d'État. Le comité de pilotage du 30 juin 2016 a entériné cet accord dans un document qui comporte les éléments suivants : les principes généraux, à savoir complémentarité, cohérence, efficience et transparence ; les principes d'organisation applicables aux modalités d'implantation et de fonctionnement des bases, ainsi qu'aux partenariats locaux principes de mise en oeuvre opérationnelle des moyens, c'est-à-dire la coordination dans l'intérêt de la personne à prendre en charge, l'emploi de l'hélicoptère le plus adapté à la mission et disponible dans les délais compatibles avec l'état du patient principes de gouvernance à l'échelon national et territorial. Par ailleurs, des indicateurs d'activité sont testés en région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre d'une expérimentation. Cela doit permettre d'objectiver et de suivre conjointement l'activité réalisée, ainsi que les éventuelles incidences de modifications des cartes d'implantation. La mission inter-inspections a salué le travail engagé par les deux directions et n'a pas recommandé la mutualisation des flottes, mais elle a soutenu l'amélioration de la coordination des moyens. Au regard de ce constat, nous sollicitons avec force le Gouvernement pour que les conclusions de l'expérimentation aboutissent le plus rapidement possible à la définition précise des principes de gouvernance à l'échelon tant national que territorial.

La problématique des déserts médicaux est, certes, cruciale, mais elle n'est pas nouvelle. Nous savons qu'il faut garantir un accès aux soins de qualité pour l'ensemble de la population, sur tout le territoire. Les enjeux sont la garantie d'un droit fondamental à la santé pour tous, mais aussi la garantie du principe de continuité du service public et du principe de l'égalité devant le service public de santé, sans oublier l'enjeu de la vitalité des territoires, notamment en zones de montagne ou rurales. À plusieurs reprises dans cet hémicycle, au cours de différents débats, nous avons souligné le manque de médecins en milieu rural. Nous nous penchons aujourd'hui sur l'aspect logistique et sur la question des transports, notamment par voie aérienne, l'hélicoptère. Nous devons toujours le garder à l'esprit : ce n'est pas au milieu rural de s'adapter à l'offre de soins ; c'est à l'offre de soins de s'adapter au milieu rural et aux besoins des populations ; c'est à l'offre de soins de s'adapter à nos montagnes. Pour cela, l'hélicoptère constitue un atout évident, une nécessité ; c'est un Haut-Savoyard qui vous le dit, Une meilleure organisation des transferts l'hélicoptère est nécessaire. C'est l'objet de cette proposition de loi. Nous ne pouvons qu'être d'accord avec cette volonté. L'implantation des moyens aériens pour le transport sanitaire peut être améliorée. Le texte initial d'Alain Bertrand, de Jacques Mézard et des membres du groupe du RDSE visait à mettre en place une stratégie nationale d'utilisation du transport sanitaire héliporté, déclinée à l'échelon régional par les agences régionales de santé.

après un état des flottes d'hélicoptères dédiées aux missions de service public. L'objectif était de déterminer le budget annuel des hélicoptères étatiques et privés, afin de rationaliser le maillage sur le territoire, mais également de réduire les coûts. Comme l'ont mentionné les orateurs précédents, il convient de distinguer le transfert primaire, qui consiste en la prise en charge des personnes pour les transporter vers les services d'urgence, du transfert secondaire, soit un transfert programmé entre établissements de santé pour une prise en charge adéquate du patient.

entre le transfert primaire et le transfert secondaire, pour lequel la durée du temps de parcours n'est pas pertinente. La rédaction initiale de la proposition de loi, qui prévoyait la gestion des transports sanitaires héliportés par les agences régionales de santé, conduisait à transférer une part importante des hélicoptères de la sécurité civile aux SAMU ; selon le rapporteur, c'était difficilement acceptable sur le terrain. Ce texte ne répondait pas à l'objectif des trente minutes et semblait trop contraignant par rapport à la régionalisation. Il aurait impliqué la mutualisation des hélicoptères des SAMU et des appareils de la sécurité civile gérés par les ARS et dont l'utilisation est déclenchée par le médecin régulateur. Or il convient de s'interroger sur les moyens pour l'ARS d'avoir autorité sur les appareils de la sécurité civile lorsque ceux-ci concourraient à des missions de police ou à des entraînements, soit 25 % de leurs vols. Qu'adviendrait-il de la continuité du service public durant ces périodes d'absence ? Le nouvel article unique, adopté en commission, prévoit donc deux principes : d'une part, une gestion mutualisée des hélicoptères susceptibles d'assurer le transport sanitaire, par un service placé auprès du Premier ministre, afin de garantir leur répartition équitable sur le territoire d'autre part, une gestion territoriale coordonnée avec celle des transports sanitaires terrestres, ainsi que la compétence du médecin régulateur pour décider de la nécessité d'un transport sanitaire héliporté. Le groupe Les Républicains est favorable au texte ainsi rédigé. Ses membres voteront donc en faveur de cette proposition de loi.

privé, il n'est aujourd'hui pas possible d'avoir recours à des moyens utiles, comme les jumelles de vision nocturne ou encore le treuillage. Ces moyens sont uniquement utilisés dans le service public, la gendarmerie et la sécurité civile. Avec le développement actuel et l'opérationnalité des services, il serait bien de fournir ces moyens au cela simplifierait de nombreux secours. Ce sont des savoir-faire que les sociétés maîtrisent du fait des qualifications de leurs pilotes et des missions de secours à personne en montagne. De tels outils sont mis à leur disposition dans des pays voisins, comme la Suisse, depuis 1990, ainsi que l'Italie ou l'Autriche. Il est regrettable qu'ils ne soient pas exploités en France.

dit assez clairement que beaucoup reste à faire si l'on entend vraiment déployer au mieux les potentialités de notre service public du secours à personne, lequel ne manque pas d'atouts. Les maux dont il souffre sont d'abord l'imparfaite coordination des responsabilités entre des acteurs multiples, aux moyens financiers divers et, surtout, encore trop enfermés dans des logiques institutionnelles trop souvent élevées au rang de « culture en juger par l'intervention de Mme la secrétaire d'État, ces acteurs ont de solides appuis au plus haut niveau ... Constatons notamment l'absence de liens institutionnels forts- les concertations ne sont pas des « liens institutionnels forts » -entre les trois principaux acteurs

Je reste à la disposition de ceux qui en douteraient. On comprend donc que la proposition de confier la gestion des secours héliportés à un « service placé auprès du Premier ministre » intégrant l'ensemble des parties prenantes ne pouvait que nous satisfaire. Elle rejoint en effet, sur une question particulière, notre proposition générale d'instituer auprès du Premier ministre une « autorité responsable de l'application du référentiel portant sur l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente Même à propos des seuls moyens héliportés, confier cette tâche au seul ministère de la santé à travers les ARS n'aurait été ni possible ni souhaitable vu le nombre d'acteurs à intervenir et, surtout, l'importance du rôle de la sécurité civile. En effet, à ce jour, les SAMU et la sécurité civile, pour ne rien dire de la gendarmerie et des douanes, disposent chacun de moyens d'intervention héliportés propres, implantés

et la nuit, ainsi que de réaliser des hélitreuillages, ce qui est rarement le cas des appareils des Héli-SMUR. Le secours à personne représente 80 % des missions de la sécurité civile.

Mettre en place une coordination entre les intervenants potentiels par une autorité extérieure aux intérêts et routines des acteurs, mais tenant compte des réalités de terrain et des solutions mises au point localement est d'autant plus nécessaire que cette autorité pourra alors décliner une doctrine globale du déploiement du service public du secours à personne garantissant qu'aucun point du territoire ne sera oublié. C'est en tout cas ainsi que j'interprète le deuxième alinéa de l'article unique de la proposition de loi : « Ce service établit les règles d'implantation des appareils afin de garantir une couverture optimale du territoire et un accès aux services

en laissant- en tout cas, je l'interprète ainsi -le soin à la régulation de décider quel est le vecteur le mieux approprié dans chaque situation particulière. Ainsi avons-nous proposé la généralisation, sur l'ensemble du territoire, de plateformes communes d'appel 15-18. Sans confondre les compétences et les responsabilités de chacun des acteurs, notamment celles des médecins régulateurs en matière de diagnostic et de soins, cela permettrait l'élaboration d'une culture commune en matière d'urgence et, surtout, l'utilisation au mieux des moyens disponibles.

Autant dire que cette proposition de loi, dont j'espère qu'elle pourra continuer sa route, vient à point pour rappeler que, dans les territoires ruraux et les îles bretonnes, l'hélicoptère reste le seul moyen permettant de répondre aux cas les plus graves, ceux pour lesquels les délais d'acheminement jusqu'au centre où ils pourront être traités sont décisifs. C'est aussi cela, « l'égalité réelle La concentration des moyens médicaux dans les villes, au nom de la qualité des plateaux techniques et de l'efficacité des soins, serait une tromperie si seuls les citadins pouvaient en bénéficier. La parole est à M. Jean-Yves Roux, pour le groupe socialiste et républicain.

: le transport sanitaire héliporté. Comme l'ont très justement fait remarquer les précédents orateurs, cette proposition de loi répond à deux enjeux majeurs, auxquels je ne peux qu'être sensible sensible : faire progresser l'accès réel à un hôpital à moins de trente minutes du lieu de prise en charge de l'urgence sanitaire ; améliorer la coordination des transports sanitaires héliportés. L'accès de la population à des soins de premiers secours en moins de trente minutes était et demeure une priorité du Gouvernement. Il s'agissait de l'un des engagements du pacte territoire-santé 1, lequel a, à ce titre, été reconduit dans le cadre du deuxième pacte territoire-santé. Je suis heureux que cet objectif, indispensable à une politique d'aménagement du territoire efficace, ait commencé à se traduire dans les faits. Je suis pour autant très attentif à ce que cet objectif puisse reposer sur un diagnostic plus précis, prenant en compte la topographie des territoires, les variations de populations, mais aussi la totalité des acteurs du transport sanitaire héliporté, disponible et formé. Le transport sanitaire héliporté revêt ainsi une signification toute particulière en montagne, en milieu rural et dans les îles. Je crois utile de le rappeler, en montagne, la distance moyenne pour accéder à un SAMU ou un SMUR est de vingt-sept kilomètres, soit contre quinze à trente-cinq minutes par hélicoptère. Certains départements, comme le mien, les Alpes-de-Haute-Provence, sont particulièrement concernés. La prise en charge de l'urgence sanitaire et l'objectif d'accessibilité à moins de trente minutes passent donc nécessairement par l'hélicoptère. Nous disposons à ce jour de nouveaux outils législatifs et réglementaires pour prendre en compte les spécificités territoriales et affiner les implantations de moyens en conséquence. L'instruction du 24 novembre 2016 relative à l'actualisation du diagnostic des populations situées à plus de trente minutes d'un accès aux soins urgents a donné aux ARS la mission d'« actualiser le diagnostic pour 2015 et 2016 des populations situées à plus de trente minutes d'un accès aux soins urgents et de mesurer les progrès effectués.

L'article 1434-3 du code de la santé publique précise que le schéma régional de santé « comporte, le cas échéant, un volet consacré aux besoins de santé spécifiques des populations des zones de montagne, notamment en termes d'accès aux soins urgents et d'évacuation des blessés, et tenant compte des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières de ces territoires. » À n'en pas douter, la stratégie nationale de transport sanitaire héliporté que les auteurs de la présente proposition de loi appellent de leurs voeux devrait tirer le plus grand bénéfice de ces diagnostics réactualisés. viens à la coordination des moyens mis en oeuvre. Je crois effectivement efficace de privilégier non une mutualisation, mais une véritable coordination, permettant d'agir en complémentarité des savoir-faire comme des équipements. À ce titre, l'ARS ne me paraît pas le seul échelon pertinent pour aboutir, en temps normal comme en temps de crise sanitaire grave, à la mise en place d'une stratégie de transport héliporté pleinement opérationnelle. Vous me permettrez, mes chers collègues, de regretter ainsi que le rôle des acteurs de la sécurité civile ne soit pas mieux identifié et n'ait pas fait l'objet d'auditions plus poussées. La sécurité civile, dont il faut louer la très grande technicité et la parfaite connaissance des territoires, est en effet indispensable à la mise en oeuvre de stratégies territoriales de transport sanitaire par hélicoptère pleinement efficientes. Les hélicoptères de la sécurité civile peuvent très bien réaliser des missions de secours à personne. Mais, inversement, les hélicoptères SAMU ne peuvent pas effectuer de missions de secours, à plus forte raison de secours complexe : durant la nuit, pendant des périodes d'intempéries météorologiques, par exemple. En effet, même si ces missions ne sont pas les plus nombreuses « quantitativement », elles sont fondamentales. Seuls les hélicoptères de la sécurité civile et de la gendarmerie peuvent les réaliser. De la même manière, la sécurité civile et l'armée sont en première ligne en cas de drame sanitaire de grande ampleur. Mon département a malheureusement été le théâtre du crash de la Germanwings qui a mobilisé, durant de nombreux jours, tous les acteurs de secours en montagne, à une très grande échelle, bouleversant aussi le recours plus quotidien au transport sanitaire héliporté. Il y a donc, je le crois, nécessité de mieux prendre en compte ces savoir-faire, comme la spécificité des flottes utilisées, dans la mise en oeuvre des futurs schémas d'implantation territoriale de transport sanitaire par hélicoptère. La coordination de deux directions, l'une relevant de l'organisation des soins, l'autre de la sécurité civile, avec, en cas de besoin, un commandement bicéphale, me paraît dans ce contexte plus pertinente. pertinente. Enfin, une plus grande efficacité de la coordination du transport sanitaire héliporté passera aussi nécessairement par un accès suffisant et itinérant à la téléphonie mobile, y compris dans les territoires les plus isolés. C'est une bataille que nous devrons mener en parallèle. La parole

est de mettre en place une stratégie nationale d'utilisation du transport sanitaire héliporté, ce qui doit permettre une prise en charge homogène, sur tout le territoire, de l'urgence sanitaire en moins de trente minutes.

est le centre de régulation où sont gérés les appels du 15, provenant d'un proche, du médecin traitant, des pompiers ou de l'ambulancier. C'est le médecin régulateur qui va, selon la gestion de l'appel, mettre en place les moyens pour prendre en charge l'urgence de la façon la plus adéquate possible pour la survie du patient. Le médecin régulateur, avec le médecin traitant ou les pompiers, dira,

Cette équipe intervient au domicile du malade ou du blessé ou va à la rencontre de l'ambulance ou du VSAB des pompiers à un endroit du trajet défini préalablement. Si le blessé ou le malade est dans un état très grave, avec des présomptions de dégradation des fonctions vitales rapide, en fonction des critères transmis, le médecin régulateur décidera d'envoyer un Héli-SMUR, service mobile d'urgence et de réanimation par hélicoptère.

sont faits entre un hôpital secondaire et un CHU pour assurer la prise en charge d'un malade dans un service spécialisé. Le transport en hélicoptère est donc bien géré par le médecin régulateur. Ce mode de transport peut être capital en zone rurale ou hyper-rurale, c'est-à-dire dans les territoires

J'ai évoqué l'emploi de l'Héli-SMUR en zone hyper-rurale, mais le cas peut aussi se présenter dans les grandes métropoles. Comment mettre en place ce transport par hélicoptère sur tout le territoire ?

que près de la moitié des hélicoptères de la sécurité civile sont en pratique employés pour des activités de transport sanitaire. Ce sont des appareils plus polyvalents

au moyen d'un service unique rattaché au Premier ministre. La gestion serait effectuée à l'échelon régional. L'objectif est le même que celui de la proposition de loi initiale : assurer un maillage territorial et garantir l'accès

loi, amendé par la commission. L'objectif est de garantir le plus vite possible la répartition équitable du transport sanitaire héliporté sur l'ensemble du territoire de la République.

Je vais mettre aux voix l'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi. Je rappelle que le vote sur l'article unique a valeur de vote sur l'ensemble de la proposition de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote ? dans le texte de la commission, l'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi visant à mettre en place une stratégie nationale d'utilisation du transport sanitaire héliporté. Merci à toutes